il faut entre 700 et 800 millions d'euros pour réparer les réseaux d'eau potable et d'assainissement en Guadeloupe. À l'époque où est née cette situation, l'État était responsable de l'affaire, avec les concessionnaires, dont Suez- c'est le nom, depuis quelque temps,

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, pour deux raisons. Sur le fond, certes, nous souscrivons bien entendu aux préoccupations de Victorin Lurel sur le réseau d'eau guadeloupéen, dont la situation est dramatique. Tout en rappelant que l'eau est une compétence décentralisée, il faut néanmoins noter que différents instruments existent d'ores et déjà, permettant d'assurer un soutien de l'État en la matière, comme le fonds exceptionnel d'investissement, qui finance des opérations dans ce domaine. Le plan de relance permettra également de financer des opérations de réfection des réseaux d'eau outre-mer. Il ne paraît donc pas pertinent de créer un programme budgétaire spécifique aux réseaux d'eau en Guadeloupe au sein de la mission « Outre-mer », alors que des dispositifs existent déjà. Par ailleurs, cet amendement est gagé sur une diminution de 40 millions d'euros des crédits du SMA, le service militaire adapté, alors que ce dernier connaît actuellement une consolidation de son mode de fonctionnement, visant notamment à assurer la transition numérique et à améliorer les taux d'encadrement.

qui commande évidemment de faire appel à la solidarité nationale pour régler le problème. Je ne reviens pas sur le plan Eau-DOM ; vous en connaissez déjà largement les contours. Il s'agit désormais d'accélérer. Votre amendement est en partie satisfait : je le vois comme un amendement d'appel-

La quasi-totalité des actions, Logement, Aménagement du territoire, Collectivités territoriales, Appui à l'accès aux financements bancaires, est en baisse. Ainsi, les crédits alloués à l'action Aménagement du territoire baissent de

Or il s'agit là d'actions prioritaires, qui, comme telles, ne sauraient faire l'objet d'économies. Cet amendement vise donc à créer un nouveau programme, « Fonds d'urgence pour l'amélioration des conditions de vie dans les outre-mer », qui serait doté de 16 millions d'euros.

Merci

avaient globalement, en 2017, un niveau de vie plus faible qu'en métropole, et les inégalités y étaient plus marquées, en particulier en Guyane, et bien plus encore à Mayotte. Le taux de pauvreté monétaire dans les DOM était deux à cinq fois plus élevé qu'en France métropolitaine. Les chômeurs, les personnes non diplômées, les jeunes et les familles monoparentales sont les plus touchés par la pauvreté. L'Insee indique en outre que la pauvreté touche un tiers de la population guadeloupéenne, quand la moitié des Guyanais et 29 % des Martiniquais vivent sous le seuil de pauvreté La vie chère est une réalité encore bien prégnante dans ces territoires. L'État reconnaît ce problème, puisqu'il octroie une « prime de vie chère » à ses fonctionnaires. Une grande partie de la population, malheureusement, ne bénéficie pas d'aide spécifique pour pallier cette différence de niveau de vie avec l'Hexagone. C'est pourquoi, en juin 2018, le Gouvernement a saisi pour avis l'Autorité de la concurrence sur le fonctionnement de la concurrence en matière d'importations et de distribution des produits de grande consommation dans les départements d'outre-mer. Il ressort de cet avis que le niveau général des prix à la consommation est plus élevé dans ces départements qu'en France métropolitaine, de 12,5 % en Guadeloupe et de 12,3 % en Martinique, notamment.

commission ? La création d'un fonds d'urgence doté de 15 millions d'euros ne me paraît pas adaptée pour lutter contre le phénomène de vie chère dans les outre-mer. Ce phénomène est structurel, et la mission comprend différents dispositifs pour le limiter, comme l'aide au fret ou l'exonération de TVA.

Le sénateur Patient a raison de rappeler que les causes de ce phénomène sont éminemment structurelles ; des questions de compétitivité, notamment, sont en jeu- je n'ai pas le temps de m'étendre ici -, des questions de fiscalité aussi : on sait très bien qu'un débat existe sur ces questions autour de l'octroi de mer ; je me suis déjà exprimé publiquement sur le sujet, je n'y reviens pas.

; de vraies questions sont posées sur les parcours de vie, le vieillissement de la population, l'existence d'un service public de bonne qualité- je ne reviens pas sur tout ce que vous avez dit, auquel je souscris parfaitement.

M. Maurice Antiste. Les producteurs agricoles des régions et collectivités d'outre-mer ont démontré durant toute l'année 2020 que la production locale joue un rôle essentiel dans nos territoires ; ils ont en effet continué à approvisionner nos populations en viandes, fruits et légumes

production locale forte, le Gouvernement peine depuis plus d'un an à répondre à la demande de revalorisation des fonds du CIOM qui émane des filières. Pourtant, le Président de la République, lors de sa visite à La Réunion, au mois d'octobre 2019, avait annoncé la préservation du fonds CIOM, ainsi que sa revalorisation.

La mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales » ne prévoit que 43 millions d'euros pour le fonds CIOM en 2021, ce qui est clairement insuffisant au regard de la situation actuelle. C'est pourquoi, en addition des 3 millions d'euros qui semblent avoir été ajoutés aux fonds CIOM, il est nécessaire de soutenir les exploitants agricoles bénéficiaires de ce fonds, en augmentant les crédits de 5 millions d'euros supplémentaires. Cet amendement vise ainsi à prélever 5 millions d'euros du programme 123, dans son action n° 09, et de les orienter vers un nouveau programme intitulé « Développement endogène des filières agricoles de diversification ». L'amendement

n'a jamais été augmenté. On nous avait assuré à l'époque qu'il n'y aurait pas de stabilisateurs budgétaires. Or ils existent depuis un moment. Cela signifie que la production agricole, notamment de diversification et d'élevage, est dans un régime malthusien :

il ne paraît pas pertinent de créer un programme budgétaire spécifique au développement endogène des filières agricoles de diversification au sein de la mission « Outre-mer », puisque cette politique publique relève principalement de la mission « Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Dominique Théophile. Cet amendement vise à mettre en place, sous la forme d'un fonds de dotation et à titre expérimental, un instrument financier qui permette au secteur de l'innovation de changer d'échelle. Les territoires ultramarins souffrent en effet d'une exiguïté qui peut entraver le développement commercial de leurs entreprises. Ce fonds doit ainsi permettre aux entreprises ultramarines de prospecter et de s'installer dans d'autres territoires ultramarins du même bassin régional, mais aussi dans l'Hexagone. ainsi d'abonder ce fonds de dotation en transférant 5 millions en autorisations d'engagement et en crédits de paiement de l'action Aménagement du territoire, du programme « Conditions de vie outre-mer », vers l'action Soutien aux entreprises, du programme « Emploi outre-mer

L'action n° 01 du programme 138 prévoit, par exemple, une dotation à hauteur de 4 millions d'euros affectée à un dispositif d'appels à projets et d'appels à manifestation d'intérêt, afin de décliner une offre spécifique pour l'émergence en outre-mer de projets innovants et environnementaux-compatibles. Monsieur le ministre,

est à M. Maurice Antiste. L'actuel projet de loi de finances fait l'impasse sur un problème majeur pour les outre-mer : les féminicides et les violences contre les femmes.

aux territoires ultramarins pour lutter contre les violences faites aux femmes. Ce fonds serait doté de 5 millions d'euros et aurait pour vocation d'accompagner les femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants à charge, en les aidant dans la poursuite de leurs activités scolaires et professionnelles, en leur rassurant un logement et en leur apportant une aide dans leurs démarches administratives et judiciaires.

Nous souscrivons bien évidemment pleinement aux préoccupations des auteurs de ces deux amendements, mais nous émettrons un avis défavorable, car la mission « Outre-mer » comporte déjà des crédits destinés à la lutte contre ce phénomène. L'action n° 04 du programme 123, qui ne porte pas de dispositifs en propre de lutte contre les inégalités, contribue à réduire les inégalités de traitement entre les femmes et les hommes au travers de subventions versées à des associations pour des projets- vingt-sept en 2019 en 2019 -relatifs, notamment, aux violences faites aux femmes, à l'égalité entre les femmes et les hommes, ainsi qu'à la lutte contre les discriminations. Il est à noter que le ministère des outre-mer, en lien avec le service des droits des femmes et de l'égalité, s'est mobilisé pour étendre l'enquête violences et rapports de genre, l'enquête afin d'actualiser les connaissances scientifiques sur la prévalence des violences dans les territoires ultramarins et d'évaluer les conséquences des violences subies par les femmes.

les établissements de santé doivent faire face à des déficits d'équipement ou à l'inexistence de spécialités. Le recours aux évacuations sanitaires, qui permettent aux patients en situation d'urgence ou nécessitant une prise en charge par un spécialiste absent du territoire de se faire soigner dans un autre territoire français ou à l'étranger, est donc nécessaire. À titre d'exemple, la Martinique ne dispose pas d'un cyclotron pour le diagnostic et le suivi des cancers. Pour Mayotte, ceux-ci sont effectués à La Réunion. C'est aussi le cas à Wallis-et-Futuna, etc. L'insularité et l'absence de certaines spécialités médicales ou chirurgicales outre-mer suscitent dès lors un nombre élevé d'évacuations sanitaires, généralement par voie aérienne. Dans le cadre de la continuité territoriale, une possibilité de prise en charge totale a été instituée, afin de permettre l'accompagnement des personnes malades devant se faire soigner. Cependant, pour les patients et leurs proches, l'éloignement lors des prises en charge, parfois longues et effectuées en dehors de leur terre d'attache, entraîne de lourdes conséquences. Afin de pallier cette difficulté et d'améliorer le système, il est proposé d'augmenter les moyens de l'action n° 03 du programme 123, en ponctionnant l'action n° 04, Financement de l'économie, du programme 138, « Emploi outre-mer ». Quel est l'avis de la commission ? Nous

nécessiterait une modification du code des transports.

ce genre de circonstances revient aux collectivités territoriales, notamment à la collectivité territoriale chef de file, le conseil départemental ou, le cas échéant, au conseil territorial en cas de fusion des deux collectivités. Je demande donc le retrait

Antiste que nous avons mis en place un dispositif à La Réunion : la caisse générale de la sécurité sociale prend en charge le billet d'avion du malade et du médecin accompagnant. Quand nous n'avons pas besoin du médecin, la caisse peut effectivement prendre en charge, lorsqu'il s'agit des mineurs, le billet

autant de dépenses sociales que l'État et la République assument. Il convient de travailler en étroite collaboration avec les différents ministères pour mettre en place de vrais moyens.

Un cluster « tourisme des outre-mer », porté conjointement par le ministère des outre-mer et Atout France, contribue à la promotion des destinations ultramarines à l'étranger par des actions communes de marketing et de communication à destination du grand public, menées par des professionnels du tourisme

est à M. Maurice Antiste. Notre amendement vise à interpeller le Gouvernement sur la situation budgétaire particulièrement préoccupante des communes ultramarines. Notre collègue Georges Patient

Ces difficultés sont la traduction d'une rigidité budgétaire qui entraîne une faible capacité d'autofinancement. Ainsi, la prise en compte de la situation des collectivités territoriales d'outre-mer doit sortir de la logique de « gestion de crise », pour favoriser un suivi plus régulier, fondé sur des données fiables et partagées par tous. Par ailleurs, il est indispensable de mieux intégrer les intérêts des outre-mer dans la construction des réformes nationales relatives aux finances locales. le déploiement d'une base statistique spécifique pour les collectivités d'outre-mer paraît incontournable. C'est pourquoi notre amendement vise à créer un observatoire des finances locales outre-mer, qui aurait pour mission la collecte, l'exploitation et la diffusion des informations statistiques et comptables en matière de finances des collectivités ultramarines. Cette structure pourrait être rattachée au comité des finances locales, le comme le propose le rapport Patient-Cazeneuve, sur le modèle de l'Observatoire des finances et de la gestion publique locales l'OFGL. Pour ce faire, il est donc proposé

On ne peut manquer de rappeler que le dispositif, en l'état, est inopérant en raison des conditions d'éligibilité. Par exemple, sur une trentaine de demandes, seules deux ont été satisfaites. Il convient ici, d'une part, de relever, le plafond des ressources, qui s'élève aujourd'hui à 6 000 euros, pour le porter à 12 000 euros, et, d'autre part, de réformer les conditions de résidence, qui ne permettent pas à un Ultramarin résidant dans l'Hexagone depuis plusieurs années de bénéficier du dispositif. Le présent amendement tend donc à abonder à hauteur de 1 million d'euros l'action n° Continuité territoriale, du programme 123, « Conditions de vie outre-mer », et à prélever du même montant l'action n° 04, Financement de l'économie, du programme 138, « Emploi outre-mer

de renforcer l'aide à la continuité funéraire. Cet amendement n'est toutefois pas plus opérant que le précédent. En effet, les conditions d'octroi de l'aide à la continuité funéraire sont fixées par le code des transports. Nous examinerons dans quelques instants un dispositif améliorant les conditions d'octroi de cette aide.

en fin d'exercice d'une proportion substantielle de l'exécution des dépenses, ce qui obère la capacité des acteurs de la chaîne de dépenses d'effectuer des redéploiements significatifs en cours d'exercice. Afin de mieux anticiper cette difficulté, un rapport sur les modalités de pilotage du programme a été remis par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel. » Un autre rapport a été remis,

les DEAL, pour donner des moyens d'ingénierie. Elle accompagnera la mise en place dans chaque territoire d'un observatoire local du logement et de l'habitat, tout en soutenant les initiatives d'adaptation des normes de construction. S'agissant, plus largement, des sous-consommations, cette question pourrait faire l'objet d'une mission au Sénat ou d'une demande d'information à la Cour des comptes de la part de la commission des finances.

On ne peut pas autoriser

affaire qui a été judiciarisée a reçu un premier résultat : l'USH a été condamnée pour avoir expulsé l'Ushom du local qu'elle louait ; vous le savez tous.

autant. Nous allons procéder au vote des crédits de la mission « Défense », figurant à l'état B. Je n'ai été saisi d'aucune demande d'explication de vote avant l'expiration du délai limite.

Le dispositif actuel permet de financer partiellement, et sous conditions de ressources, le billet d'avion pour assister aux obsèques d'un parent, d'un enfant ou d'un conjoint en outre-mer, lorsque le bénéficiaire réside en métropole. Cette mesure, bien qu'elle soit salutaire, demeure lacunaire, en ce qu'elle s'adapte peu aux réalités familiales et aux besoins de mobilité des Français d'outre-mer. C'est pourquoi nous souhaitons, par le présent amendement, clarifier la possibilité de se rendre au chevet du proche en fin de vie, ouvrir le dispositif aux frères et soeurs et étendre l'éligibilité de ce dispositif tant aux déplacements entre les collectivités d'outre-mer qu'aux déplacements entre Selon les estimations du Gouvernement, cette mesure concernerait 317 déplacements par an, pour un montant de 100 000 euros, sur un budget total de 6 millions d'euros.

des 256 000 habitants de l'île y est née, le reste de la population venant surtout des Comores : comme le dit notre éminent collègue Mansour Kamardine, député de Mayotte, plus de 40 % de la population est désormais clandestine. De telles circonstances pèsent lourdement sur la situation démographique, économique et sociale du département. Le déséquilibre s'est encore accru entre 2012 et 2017 : ainsi, le déficit migratoire des natifs de Mayotte a presque doublé par rapport à la période 2007-2012, notamment du fait des départs

Ainsi, le nombre de demandeurs d'asile en provenance d'Afrique est passé de moins de 100, en 2014, à plus de 1000 cette année. Mayotte est en train de devenir une nouvelle voie d'accès vers l'Europe. Même si ce sujet relève plus précisément de la mission « Immigration, asile et intégration », nous devons nous interroger sur la part sociale en matière migratoire. Je sais que le Sénat s'oppose systématiquement aux amendements demandant des rapports, mais je crois que nous devons ouvrir le débat : si nous demandons de tels documents, c'est justement parce que le Gouvernement, interrogé à plusieurs reprises, n'a jamais répondu précisément à ces questions, en dépit de toutes nos sollicitations.

Même si l'aide médicale d'État n'est pas applicable à Mayotte, les étrangers en situation irrégulière peuvent s'y faire soigner dans le centre hospitalier ou en ville, pour un montant qui demeure aujourd'hui inconnu.

commission ? J'émets un avis défavorable, par cohérence avec la position de principe de la commission des finances sur les rapports parlementaires.

de la réforme de la rémunération qui a été engagée et qui semble porter ses fruits, puisque les recrutements, malgré un contexte sanitaire difficile, se sont plutôt bien effectués.

et l'effort budgétaire qui l'accompagnait avaient pour objectif de compenser une perte de matériels ! L'objectif annoncé et voté était bien d'améliorer le contrat opérationnel, ainsi que la disponibilité. Enfin, on nous annonce qu'il est possible d'acquérir, non plus 12 Rafale, mais moins,

La décision est imminente, nous dit-on, mais elle tarde cependant à se manifester. Je ne puis croire qu'un enjeu aussi fondamental soit dépendant du calendrier de communication présidentiel ! Qu'en est-il

comme si c'était l'alpha et l'oméga, comme si la menace pouvait se calculer en PIB ... Il s'agit simplement de mesurer un effort financier. Je m'inquiète que, avec une chute probable du PIB, nous n'atteignions malgré nous très vite les 2 %. Déjà, une petite musique se fait jour en ce sens

Deuxièmement, le produit de la vente des Rafale reviendra-t-il bien intégralement au ministère ? Troisièmement, pouvez-vous vous engager sur le fait que la vente des Rafale ne se traduira pas par une révision à la baisse du contrat opérationnel ? Quatrièmement, quand sera annoncé officiellement le choix de la propulsion du porte-avions ? Cinquièmement, et enfin, la baisse probable du PIB est-elle de nature à remettre en cause l'enveloppe globale en valeur absolue de la loi de programmation

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le programme 144 voit ses crédits progresser de 8,9 %. Ces crédits commenceront en 2021 à financer le nouveau fonds innovation défense, le FID ; d'après ce que nous avons compris, sa montée en puissance se fera sur cinq ans.

des éléments factuels incitant les banques à la prudence : je pense en particulier aux sanctions extraterritoriales américaines, qui avaient frappé BNP Paribas

à ce stade, madame la ministre, que pour faire évoluer la situation, il faudrait agir dans trois dimensions : établir un réel dialogue autour des représentants de l'État, entre les entreprises de la BITD et les banques ; faire comprendre, au-delà de la communauté de défense, la relation directe entre l'existence de la BITD et la souveraineté nationale ; oeuvrer à défendre notre souveraineté économique. C'est un vaste sujet, que nous ne réglerons pas lors de ce débat. Enfin, je voudrais signaler que nous avons été étonnés, pour ne pas dire choqués, de découvrir la réduction de voilure de notre réseau de missions militaires à l'étranger, dans des postes pourtant très sensibles : Alger, Tunis, Amman, Tbilissi- ce poste couvre l'Arménie et l'Azerbaïdjan -, et même Londres et Moscou

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le programme 144 porte une partie des crédits du renseignement pour un peu plus de 400 millions d'euros. Il concerne deux services du premier cercle, qui dépendent du ministère des armées : la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) et la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD).

Dans le programme 144, ses crédits s'établiront en 2021 à 388 millions d'euros, soit une hausse de 11,4 %. Cette augmentation notable traduit la poursuite d'un effort d'investissement Il s'agit, d'une part, de mettre le parc immobilier à niveau, à la fois pour faire face à la croissance des effectifs et pour rénover certains bâtiments vétustes, d'autre part, d'accroître les capacités les capacités techniques, en particulier dans des domaines où le progrès technologique impose des investissements soutenus pour qu'ils soient maintenus à un bon niveau. Il faut savoir que les capacités techniques de la DGSE ont vocation à être partagées avec les cinq autres services du premier cercle. de la situation de la DGSE, il convient d'examiner aussi ses moyens humains. La DGSE compte aujourd'hui environ 7 100 personnes. Ses effectifs devraient rester stables l'an prochain, avant de reprendre leur progression pour atteindre 7 800 agents en 2025. En intégrant les dépenses de personnel, les crédits de la DGSE s'établiront en 2021 à 880 millions d'euros, soit une hausse de 7,7 %. Enfin, mentionnons également l'existence des fonds spéciaux. La part principale des 76,4 millions d'euros de fonds spéciaux va à la DGSE. Pour porter une appréciation sur ce niveau de crédit, il faut considérer néanmoins que l'effort financier de la France dans le domaine du renseignement extérieur reste sans doute encore un peu inférieur à celui de l'Allemagne et très sensiblement inférieur à celui du Royaume-Uni. et de la sécurité de la défense, un service en transformation qui réoriente de plus en plus son activité sur le renseignement. Rappelons que, avec 1 500 agents, ce service doit mener un nombre très élevé d'enquêtes administratives- 311 000 l'année passée -en vue d'assurer globalement la protection de nos forces. La DRSD a donc dû beaucoup se moderniser et mettre en place des outils d'aide au traitement des dossiers en recourant notamment, et de plus en plus, à l'intelligence artificielle. Ses crédits inscrits dans le programme 144 progresseront de 12,2 %. En y incluant les dépenses de personnel, les crédits du service s'établiront à 143,2 millions d'euros.

Or l'amélioration de l'activité opérationnelle n'apparaît pas comme une priorité du budget, contrairement à l'entretien programmé des matériels (EPM), qui bénéficie en 2021 de 39 % des crédits du programme, soit 4,12 milliards d'euros.

la situation de l'activité opérationnelle et de la disponibilité technique opérationnelle (DTO) n'est pas satisfaisante. La remontée de l'activité opérationnelle aux normes d'activité de l'OTAN a été repoussée à 2025. à 2025. Nos soldats ne sont donc pas assez entraînés par rapport aux normes internationales et ne le seront pas avant 2025. Cela n'est plus compatible avec le constat que nous faisons de la multiplication et du durcissement des conflits. Deuxième constat : les capacités industrielles des acteurs chargés de la maintenance et de leurs sous-traitants doivent faire l'objet d'une grande vigilance. Troisième constat : les crédits consacrés à l'entretien programmé du matériel devaient s'établir à 4,4 milliards d'euros par an.

tels que le coût de réparation de la Perle pour 70 millions d'euros, le surcoût lié à l'utilisation d'aéronefs vieillissants ou la livraison des 12 Rafale destinés à la Grèce. D'autres facteurs sont structurels et découlent de la mise en oeuvre de la politique de verticalisation des contrats d'EPM, notamment dans le domaine aéronautique. Ces contrats verticalisés se traduisent paradoxalement, dans un premier temps, par des surcoûts mise en oeuvre de nouvelles chaînes industrielles d'EPM, remise à niveau des stocks de pièces de rechange étatiques transférées lors de la mise en oeuvre du contrat verticalisé à l'industriel. Tous ces facteurs s'ajoutent à la projection de nos troupes sur de multiples théâtres d'opérations extérieures et à la sur-exécution des contrats opérationnels, qui avait conduit à l'inscription de 500 millions d'euros supplémentaires pour les deux dernières annuités de la précédente LPM.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le modèle de soutien des forces armées a souffert du double effet de la révision générale des politiques publiques et de la précédente loi relative à la programmation militaire pour La commission a d'ailleurs souligné le décalage entre moyens alloués et impératifs d'efficacité, dans un contexte de haute intensité sanitaire. du commissariat des armées (SCA) a perdu 30 % de ses effectifs au cours des six dernières années. Nous veillerons tout au long de l'exécution de la LPM à ce que la direction centrale ne soit pas de nouveau confrontée à une pénurie de moyens humains, comme ce fut le cas lors de la précédente période de programmation. De même, la professionnalisation des filières du SCA dépend de sa capacité à bâtir des parcours et des carrières. Le niveau de qualification des personnels affectés par les armées au SCA doit correspondre plus systématiquement aux profils des postes.

La mise en oeuvre du nouveau modèle hospitalier militaire sera l'un des axes de la stratégie SSA 2030 qui est en cours de définition. Les cartes ont été rebattues par la pandémie. Les huit hôpitaux d'instruction des armées participent à l'offre de soins à l'échelle d'un territoire. À cet égard, les élus locaux doivent être étroitement associés à la définition de cette offre de soins. difficulté du SSA concerne la médecine des forces. Faute d'effectifs suffisants, les mêmes personnels supportent la charge de projection en OPEX. Le taux de projection des équipes médicales est supérieur à 100 %, malgré l'apport des réservistes et il atteint 200 % pour les équipes chirurgicales. Cette sursollicitation nuit à la fidélisation des personnels. Les conclusions du Ségur de la santé pèseront sur l'attractivité du SSA et devront sans doute être compensées dans le cadre de l'actualisation de la loi de programmation militaire. Enfin, la vaccination contre la covid en France ne sera peut-être pas intégrée aux recommandations vaccinales adressées aux militaires. les militaires embarqués ou déployés en OPEX doivent absolument bénéficier de mesures de protection adéquates face à la pandémie. Je souhaiterais entendre Mme la ministre sur ce sujet sensible pour la commission des

des pensions sont particulières : liquidation possible au bout de vingt-sept ans pour les officiers de carrière, de dix-sept ans pour les non-officiers, liquidation sans décote deux ans plus tard, durée de cotisation sensiblement majorée par des bonifications spécifiques. Ce système encourage les reconversions en milieu de carrière et sert une démographie qui doit s'accorder avec la « haute intensité ». Or, du fait des réformes paramétriques successives, l'âge moyen des militaires s'est accru de près de trois ans jusqu'en 2016, que la croissance des effectifs ne stoppe ce vieillissement. Toutefois, des entrées plus tardives sur le marché du travail et l'effet du chômage sur les reconversions incitent à la prudence. Dans le système à points envisagé par le Gouvernement, les primes seraient prises en compte.

et sont en cours de refonte -, ainsi que du profil de carrière, plus ou moins ascendant. Les modalités des réversions seraient aussi à surveiller. Dans ce contexte, les pensions suscitent une inquiétude chez les militaires. C'est la raison pour laquelle la commission continuera à exercer son devoir de vigilance et que nous serons certainement amenés à creuser par la suite. Je me suis par ailleurs intéressé aux méthodes de recrutement de l'armée de terre, à la fois innovantes et prometteuses. Elles misent sur le et l'intelligence artificielle pour repérer sur les réseaux sociaux les profils pertinents et leur adresser messages

avis. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi de finances pour 2021 suit le trait voulu par le Président de la République et par vous, madame la ministre, à travers la loi de programmation militaire.

plein, les armées ont été réactives et ont mis en place des innovations afin d'atteindre les objectifs, comme le maintien en service au-delà des limites d'âge, le maintien de la durée du service ou du contrat, le réengagement d'anciens militaires, l'anticipation du recrutement de contractuels ou l'assouplissement

dans le contexte de la crise sanitaire, l'armée a su s'adapter à l'urgence- nous l'indiquons dans le rapport pour avis. Ainsi, pour l'ensemble du ministère, le schéma d'emploi perdrait 112 emplois en 2020 sur les 300 équivalents temps plein

des recrutements. Depuis 2014, on assiste de manière régulière à une dégradation de la qualité des viviers et à une augmentation de l'attrition.

2021 doit être celle de l'actualisation de la loi de programmation militaire. Cette actualisation devra consolider la programmation : ce n'est que dans la durée, d'ici à 2030, que la LPM actuelle et la suivante produiront tous leurs effets.

Pour l'armée de terre, les deux tiers du programme Scorpion restent à contractualiser. L'effort sur les équipements « à hauteur d'homme » doit se poursuivre. Pour la marine, il est urgent de lancer le porte-avions de nouvelle génération. À cet égard, la commission préconise une propulsion nucléaire, mais la décision présidentielle est attendue depuis maintenant près d'un an.

Nous le ressentons tous, madame la ministre, je tenais à vous le dire avec la plus grande sincérité. Il n'est pas concevable que la trajectoire financière et, donc, les ambitions de la politique de défense puissent être demain révisées en dehors de tout contrôle parlementaire. Madame la ministre, nous confirmez-vous, comme vous l'a déjà demandé le rapporteur spécial, que la voie législative est bien celle qu'a retenue le Gouvernement ? J'en viens au contrat d'exportation du Rafale en cours de négociation avec la Grèce, qui conduit à prélever 12 avions sur nos forces et à décaler de plusieurs mois les livraisons à l'armée de l'air à l'armée de l'air d'appareils neufs prévues à partir de 2022. Nous craignons des conséquences opérationnelles, voire un effet déstructurant si l'opération devait se renouveler avec la Croatie, ce que nous espérons par ailleurs. L'exportation du Rafale est évidemment une bonne nouvelle. Ce pari de la LPM, qui est en passe d'être tenu, permettra, je le rappelle, de maintenir en activité les chaînes de production.

Les montants sont en cours de négociation, non seulement pour les appareils eux-mêmes, mais aussi pour les capteurs et l'ensemble du matériel qui sera cédé. La somme de 600 millions d'euros est évoquée. Celle-ci sera évidemment loin d'être suffisante pour financer l'acquisition d'avions et d'équipements neufs. Il manque plusieurs centaines de millions d'euros. Comment dégagerez-vous les crédits nécessaires, madame la ministre, alors que les budgets sont déjà conçus au plus juste ? Nos armées, nos industriels ont besoin de perspectives de long terme, encore plus en cette année de crise

risque fort de poser un problème de disponibilité des avions pour l'armée de l'air et de l'espace dans les cinq ans à venir sans anticipation de notre part dès à présent. En effet, même s'ils étaient commandés aujourd'hui, les avions neufs ne seraient pas livrés avant 2025. Or, madame la ministre, vous nous avez annoncé il y a quelques semaines la commande de douze appareils neufs. La commande grecque a été annoncée au mois de septembre dernier, nous sommes au début du mois de décembre : quand ces contrats seront-ils finalisés ? Nous confirmez-vous que les commandes seront passées avant la fin de l'année ?

Madame la ministre, étant donné le rôle des parlementaires allemands, le Gouvernement n'a-t-il pas intérêt à compter davantage sur la diplomatie parlementaire française en associant les parlementaires au dialogue franco-allemand ? Pouvez-vous également nous donner quelques informations sur les négociations avec notre partenaire espagnol et sur la place qui lui est réservée dans le programme SCAF ? Enfin, le plan de relance de la fin de l'été ignore la base industrielle et technologique de défense. À titre de comparaison, nos voisins britanniques ont pris des mesures fortes : le Premier ministre Boris Johnson a récemment annoncé un effort massif en faveur de la défense, dont le budget augmentera de 27 milliards d'euros en quatre ans, soit 18 milliards d'euros de plus que prévu. Ce montant est à comparer aux 600 millions d'euros de commandes que le ministère des armées s'est engagé à passer dans le cadre du plan de soutien à l'aéronautique. L'investissement britannique risque fort d'accélérer le programme , dont dont le lancement est prévu en 2035, soit cinq ans avant l'achèvement du programme SCAF. Devrions-nous être plus attentifs à ce programme, potentiellement concurrent ? En tout cas, c'est une raison supplémentaire de regretter que la défense ne bénéficie pas du plan de relance, qui aurait pu très utilement renforcer la LPM. Mes chers Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, dans une situation économique et financière compliquée, préserver et renforcer l'état de nos fonctions régaliennes est fondamental pour garder la main sur notre destinée nationale, notre autonomie stratégique et notre souveraineté.

l'augmentation de 3,3 % des crédits du programme 178 ne prend pas en compte le surcoût des opérations intérieures de 30 millions d'euros, résultat d'une situation sécuritaire explosive dans notre pays. Le surcoût des OPEX et des missions intérieures s'élève à 1,4 milliard d'euros. Si tous les ministères ne prennent pas leur part dans ce surcoût, conformément à ce que prévoit la loi de programmation militaire, ce sont nos armées, les hommes et les femmes qui les composent, la réparation et la modernisation des équipements qui en subiront les conséquences. Sur les quatorze indicateurs d'activité opérationnelle, un seul devrait être conforme aux normes de l'OTAN en 2021, pour nos armées de terre, de l'air et de l'espace et notre marine nationale, à l'heure où la Turquie attise les tensions non seulement en Arménie et en Libye, mais aussi en Grèce, à Chypre et en Méditerranée. Le chef d'état-major de l'armée de terre en a fait sa priorité, « être prêt à la haute intensité », mais le Gouvernement ne lui donne pas les moyens de disposer d'équipements à la hauteur, des entraînements adaptés, d'une industrie de soutien.

des efforts consentis par nos voisins allemands et britanniques. De la même manière, l'augmentation de 10 % des crédits alloués à la base industrielle de technologie et de défense est une dépense publique en pure perte si l'État ne soutient pas ses entreprises de défense. Ces

Je ne vous cache pas que, en cette période de disette budgétaire, les priorités d'action du Gouvernement, essentiellement tournées vers le régalien, ont de quoi susciter des interrogations. Le traitement de la crise n'est pas identique dans les différents ministères. Contrairement à nos homologues allemands ou américains, les parlementaires que nous sommes sont impuissants à déterminer la stratégie de défense française, notamment en ce qui concerne les opérations extérieures. Notre rôle revient essentiellement à signer un chèque quand vous nous présentez la facture, sur laquelle nous n'avons pas notre mot à dire.

matérielles de vie. Or ce n'est pas tout à fait le cas : les deux tiers des montants ouverts en autorisations d'engagement sont dédiés à l'équipement des forces et un tiers seulement est consacré aux dépenses de personnel. Finalement, il reste moins de 1 milliard d'euros pour soutenir matériellement les femmes et les hommes qui servent la France. Nous sommes donc loin du budget « à hauteur d'homme » que vous aviez annoncé, madame la ministre.

Vous l'aurez compris, même si je salue l'augmentation des crédits alloués à l'action Contrôle général des armées, je pense qu'elle est encore insuffisante pour véritablement démocratiser des outils comme la plateforme Thémis. Au-delà de la dimension humaine, la cohésion au sein des armées est essentielle d'un point de vue stratégique. Un budget « à hauteur d'homme » doit aussi permettre d'améliorer les conditions de vie matérielle des soldats.

En parlant de rénovation énergétique, nous saluons l'effort entrepris pour diminuer la consommation d'énergie de nos armées. J'ai cru relever que vous visiez l'éradication des chaudières au fioul et au charbon d'ici à 2031. Cette échéance me semble encore très lointaine, sachant que le Gouvernement a prévu, et c'est heureux, d'interdire les chaudières au fioul neuves neuves en 2022 et d'éradiquer les chaudières au fioul d'ici à 2028. Il serait souhaitable que la puissance publique ne soit pas à la traîne sur les objectifs qu'elle fixe aux particuliers et qu'au contraire elle montre l'exemple. de même pas comme si vous vous manquiez de moyens pour consacrer plus de 500 millions d'euros en six ans à l'amélioration des performances énergétique de nos armées ! Ces deux points, le mal-être et les conditions de vie de nos militaires, m'amènent à la question de la fidélisation.

Pourtant, je le répète, le mal-être et les conditions de vie que nous offrons à nos militaires sont loin d'être « à hauteur d'homme ». Les problématiques de recrutement qui en résultent sont donc logiques. une remarque d'ordre plus général : la crise que connaît l'OTAN, avec le retrait américain et les provocations de la Turquie, remet sur la table le besoin d'une Europe de la défense. Cela justifierait le maintien et le développement de notre appareil militaire, notamment de la dissuasion nucléaire double, qui n'est pas dimensionnée pour le seul besoin national.

En attendant, les puissances nucléaires modernisent leur arsenal et la perspective d'un monde sans armes nucléaires est bien lointaine. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s'abstiendra sur les crédits

permettez-moi tout d'abord d'exprimer l'honneur qui m'est fait d'intervenir pour la première fois à cette tribune et d'exprimer devant vous la position du groupe RDPI sur la mission « Défense » du projet de loi de finances pour 2021. Cette année encore, le projet de budget présenté par le Gouvernement pour la mission « Défense » est en hausse significative. Il s'élève à 39,2 milliards d'euros en crédits de paiement, soit une augmentation de 4,5 % correspondant à 1,7 milliard d'euros. Depuis la loi de finances initiale pour 2017, les crédits de la mission « Défense » ont ainsi augmenté de 22 %, soit 6,8 milliards d'euros. Nous ne pouvons que nous réjouir du respect des engagements tenus, puisque le budget 2021 est conforme à la trajectoire établie par la loi relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 du 13 juillet 2018, et ce pour la troisième année consécutive, ce qui est relativement inédit dans l'histoire de ces lois de programmation. Toutefois, si nous souhaitons extraire toute la quintessence de cette loi de programmation militaire, madame la ministre, il sera indispensable d'appliquer les différents budgets annoncés jusqu'à leur terme, sans quoi nos armées en perdront les principaux bénéfices. Cet effort exceptionnel répond aux besoins de transformation et d'adaptation de nos armées à un monde sans cesse plus instable, marqué aussi bien par l'émergence de nouvelles menaces et de nouveaux espaces de conflictualité que par une course technologique effrénée. L'effort consenti par la Nation en faveur des armées est d'autant plus remarquable qu'il s'inscrit dans un contexte budgétaire contraint en raison de la pandémie, avec les conséquences économiques et budgétaires que nous connaissons.

Le budget 2021 permet de répondre au souhait d'avoir une politique de défense humaine, ambitieuse et innovante. Humaine d'abord, car ce budget 2021 répond au besoin d'un modèle d'armée « à hauteur d'homme » complet, équilibré et soutenable dans la durée, qui affronte véritablement les défis de recrutement et de fidélisation de nos militaires, améliore les conditions d'hébergement et poursuit le renforcement des équipements d'accompagnement et de protection de nos soldats. Ambitieuse ensuite, car, avec 21 milliards d'euros en autorisations d'engagement et 13,6 milliards d'euros en crédits de paiement, le programme 146, « Équipement des forces » bénéficie de l'essentiel de cette hausse et capte une bonne partie des nouveaux crédits. Ces crédits permettront de poursuivre la remontée en puissance capacitaire de nos armées. Je signale notamment la livraison de nombreux aéronefs et matériels terrestres avec 157 blindés Griffon et 20 blindés dans le cadre du programme Scorpion, ainsi que d'une nouvelle frégate multi-missions de défense aérienne. Dans le domaine prioritaire du spatial, un satellite CSO (Composante spatiale optique) et un système de satellites Ceres (Capacité d'écoute et de renseignement électromagnétiques spatiale) seront également livrés. Innovante enfin, car une armée qui innove est une armée qui construit son autonomie stratégique. Cet élan technologique, le ministère des armées a su le saisir à plusieurs titres. À très court terme, en matière de lutte contre la covid-19, l'Agence de l'innovation de défense a investi dans des solutions innovantes pour faire face à ce coronavirus, comme le projet MakAir de développement d'un respirateur artificiel simplifié. Il prévoit le développement des armes hypersoniques et de technologies quantiques, un virage technologique qu'il convient de ne pas manquer. En matière d'investissement R&D de long terme, il a intensifié le partenariat public-privé en travaillant plus intimement avec des pépites françaises leader de domaines technologiques de pointe. Cet axe, malgré la création du fonds d'investissement Definnov, reste perfectible. En matière d'anticipation, enfin, il travaille dès à présent aux conflits du futur, à l'horizon 2030-2060. Tel est l'objet du projet ambitieux, en partenariat avec l'Agence de l'innovation de défense, ou à travers notre armée de l'air et de l'espace, avec le système de combat aérien du futur, le fameux SCAF dont le démonstrateur doit être impérativement lancé l'année prochaine. Chers collègues, nous le voyons bien, que ce soit en opérations extérieures, afin d'assurer notre souveraineté, ou sur le territoire national, nos forces armées demeurent engagées à un rythme soutenu. Je salue ici leur infaillible et infatigable abnégation. Plus que jamais, la France doit se doter d'une armée moderne et polyvalente pouvant répondre aux nombreux défis sécuritaires contemporains, mais aussi au retour potentiel des conflits à haute intensité. Ce budget, construit à partir de la réalité opérationnelle de notre engagement militaire, redonnera à nos armées les moyens d'assurer leur mission et de tracer un chemin vers notre Ambition 2030. Il démontre à nos forces armées qu'elles peuvent à leur tour compter sur nous. notre groupe est fier de soutenir votre action volontaire et ambitieuse, qui met un terme aux coupes budgétaires et autres renoncements infligés à nos armées ces vingt dernières années. La pandémie de la covid-19, mais aussi des catastrophes industrielles ou naturelles ont mis en exergue l'importance de disposer d'une capacité de réaction et de résilience à la hauteur. Ces différents événements se sont effectivement traduits, ces derniers mois, par une forte mobilisation des armées et notamment du service de santé des armées (SSA), au travers de l'opération Résilience.

Enfin, il faut en être conscient, un budget de la défense irrigue bien au-delà du simple périmètre militaire et contribuera de façon déterminante à la relance économique de la France et à la Les dépenses dédiées aux équipements sont directement injectées dans des entreprises stratégiques, notamment les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries, qui constituent l'essentiel du tissu industriel de la base industrielle et technologique de défense (BITD), composé d'environ 4 000 entreprises employant quelque 200 000 personnes. Au-delà du soutien de nos armées, ce budget est donc un plan de soutien massif à l'industrie de défense et aux emplois dans nos territoires, durement frappés par la crise. Pour toutes ces raisons, le groupe RDPI votera avec fierté en faveur de la mission « Défense ». La parole

dans le contexte de conflictualité élevé que le monde connaît actuellement, le budget de la mission « Défense » invite à la plus grande vigilance quant au maintien de ses moyens. La Revue stratégique de défense et de sécurité nationale de 2017 prenait acte du « retour des puissances » dans les relations internationales. C'est un fait, les ambitions militaires de la Chine, le réveil stratégique de la Russie et les visées conquérantes de la Turquie remettent en cause l'ordre multilatéral, alors même que notre pays est attaché à une régulation des relations internationales avant tout fondée sur le droit. Le ministre des affaires étrangères l'a rappelé ici même, la semaine dernière, à propos du Haut-Karabagh. Je n'oublie pas, bien sûr, la lutte contre le terrorisme islamiste, qui impose l'adaptation de nos forces armées et de nos services de renseignement face à une menace protéiforme. À cet égard, je salue le courage de nos soldats et leurs derniers succès obtenus dans la bande sahélo-saharienne ; je pense notamment à l'élimination d'un important chef militaire malien appartenant à la branche sahélienne d'Al-Qaïda. Cette avancée s'ajoute à d'autres, qui répondent à mon sens à la question, parfois soulevée, d'un potentiel enlisement de la force Barkhane au Sahel. Comme le disait Winston Churchill, « le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal : c'est le courage de continuer qui compte Il s'agit pour moi non pas de vanter une posture « va-t-en-guerre », mais de rappeler combien le basculement de pays du continent africain dans le giron terroriste serait coûteux pour les démocraties occidentales, en premier lieu bien sûr pour les populations locales. locales. Quelles guerres se gagnent à travers le prisme du temps court ? Peu, hélas ... Dans ces conditions difficiles, on ne peut que se réjouir de la poursuite, en 2021, d'une montée en charge des moyens budgétaires de la défense, conformément à la trajectoire tracée par la loi de programmation militaire 2019-2025, même si l'effort devrait être plus important à partir de 2023, comme l'ont fait justement remarquer les rapporteurs

Cependant, en marge de la mission, je m'inquiète de l'état de l'écosystème industriel qui lui est lié. L'industrie aéronautique est en souffrance, alors qu'elle est un fleuron de notre export et représente surtout des milliers d'emplois de PME qui irriguent nos territoires.

C'est une bonne chose, mais les livraisons seront-elles tenues, par exemple au regard de la cible de 128 blindés Griffon qui ne sera pas atteinte cette année ? Enfin, en tant que sénateur du Var, je pense aussi aux moyens de la marine nationale. Aussi, madame la ministre, je salue les efforts entrepris depuis trois ans en sa faveur. Le nouveau sous-marin Suffren et la réussite de son tir de missile de croisière illustrent la remontée en puissance et témoignent de l'effort budgétaire de plusieurs années. Il faut cependant éviter la multiplication des ruptures temporaires de capacité qu'on a pu connaître, dans un contexte de tensions politiques et criminelles croissantes en haute mer, lesquelles entraînent un haut niveau d'engagement opérationnel de nos forces navales. En marge de cette nécessité de donner à notre marine les moyens de ses missions, je me réjouis de la poursuite du plan Famille. Il est fondamental de porter une attention soutenue à la vie quotidienne de nos marins, en retour de l'abnégation que suppose leur vie à bord. Pour terminer, je profite de cette tribune pour saluer particulièrement le travail de tous les ingénieurs, techniciens et ouvriers de nos arsenaux, qu'ils soient de Brest, de Cherbourg, de Toulon,

et ils sont au rendez-vous : le renforcement de l'opération Sentinelle après les attentats, les opérations Résilience pour la crise sanitaire, l'opération Amitié pour le Liban

En cet instant, avec vous tous, j'ai une pensée pour les 35 000 hommes et femmes de nos forces armées, déployés sur le territoire national comme à l'extérieur. Cette année, je le rappelle, dix militaires français ont payé de leur vie leur engagement, et je tiens ici, en notre nom à tous, à leur rendre encore un ultime hommage. Ce sont ces soldats, ces marins, ces aviateurs, dont l'abnégation et le courage forcent l'admiration. Ils sont l'excellence de nos armées. Ce sont eux qui, si souvent, sont en première ligne, face à la dégradation du contexte stratégique.

Il continue de répandre son idéologie mortifère sur tous les continents, singulièrement en Europe. Notre pays a encore été cette année durement éprouvé. On note ensuite retour des États puissances : l'actualité ne cesse de nous en donner des exemples et, à nos portes, la Méditerranée en est le théâtre. La Turquie n'hésite plus à user de la force militaire, la Russie se place en position centrale, tandis que l'Europe paraît plus qu'hésitante, préférant bien souvent les condamnations verbales, qu'il faut âprement négocier, négocier, aux démonstrations de puissance qui ne correspondent ni à sa culture ni à l'ambition d'un certain nombre de ses membres. L'escalade récente de la violence dans le Haut-Karabagh nous montre dans quelles impasses nous conduit cette impuissance. L'élection d'un nouveau président des États-Unis changera-t-elle la donne ? Rien n'est moins sûr, car, nous le savons, les États-Unis réorienteront durablement leur effort militaire vers l'Indopacifique. Tous nos partenaires européens feraient bien de le comprendre et de continuer d'avancer dans le sens du renforcement de l'autonomie stratégique européenne. Dans ce contexte, avec 39,2 milliards d'euros, la mission « Défense » de ce projet de loi de finances, le troisième depuis l'adoption de la loi de programmation militaire, est conforme à la trajectoire prévue. Peut-on néanmoins faire comme si rien ne s'était passé au cours de l'année 2020 ? Peut-on ainsi considérer que la LPM de 2018 constitue en elle-même un plan de relance suffisant pour répondre à la grave crise, non seulement sanitaire, mais aussi économique et géopolitique, que nous traversons actuellement ? Oui, l'effort

ici. Oui, les nouveaux matériels arrivent : cette année a été notamment marquée par la livraison du nouveau sous-marin nucléaire d'attaque (SNA) Suffren après le succès de ses essais à la mer. Le premier tir de missile de croisière naval depuis ce SNA inaugure pour notre pays une nouvelle capacité stratégique, qui sera décisive pour nos armées. L'entretien programmé du matériel a bénéficié d'un effort important. Autant dire que c'était vraiment nécessaire, vu la détérioration de la disponibilité des équipements au cours de la précédente période de programmation.

Par ailleurs, comme chaque année à la même période, la fin de gestion vient un peu tempérer notre satisfaction. Le surcoût des opérations extérieures et des missions intérieures en 2020 s'est révélé une fois de plus supérieur aux montants provisionnés. Le solde s'élève à 236 millions d'euros : il est financé par des redéploiements ou des annulations de crédits, dont 124 millions d'euros prélevés sur le programme « Équipement des forces » par la loi de finances rectificative. Ce n'est pas toujours le bon signe qui nous est envoyé. signe qui nous est envoyé. Dans ce budget, une fois de plus, il semble que l'on ignore l'article 4 de la LPM, qui prévoit une solidarité interministérielle pour le financement de ce surcoût ; nous le déplorons.

Vous avez pu entendre à travers les interventions de nos rapporteurs une inquiétude, parce que la crise économique est une bombe à retardement pour notre industrie de défense. Les carnets de commandes passés ont masqué la crise en 2020, mais les prochaines années risquent d'être dévastatrices.

malgré tout rassurer, même si ce n'est pas toujours le sentiment de nos industriels. L'aéronautique a bénéficié d'un plan de soutien, mais aucune mesure spécifique n'a été prise à l'intention des industries terrestres et navales. Nous tenons à vous faire part de leur inquiétude. Chacun connaît pourtant le potentiel de la BITD : ce sont 200 000 emplois de haute technologie, non délocalisables, des milliers de PME irriguant nos territoires. C'est un secteur capable de transformer rapidement la commande publique en croissance, en emplois et en recettes fiscales. Dès lors, pourquoi s'en priver, alors que l'économie connaît une récession exceptionnelle par son ampleur et que les besoins en matière de défense restent criants ?

Faites en sorte que nous ne soyons pas mis devant le fait accompli, face à des arbitrages opaques sur lesquels les parlementaires n'auraient aucun droit de regard. Vous savez le soutien que le Parlement vous a apporté pour la LPM, il en sera de même pour son actualisation. Il va de soi que seule une loi peut modifier, compléter ou actualiser une loi. L'actualisation de la LPM devra être un rendez-vous de transparence démocratique, car ses enjeux sont essentiels. Chaque euro comptera. De grands programmes doivent être sanctuarisés : le système de combat aérien du futur, le char du futur, le porte-avions de nouvelle génération. Des questions restent en suspens et nous devrons en débattre. Au-delà de ces programmes phares, au-delà du renouvellement indispensable de notre dissuasion nucléaire, c'est bien notre modèle d'armée complet, gage de notre souveraineté, qui est en jeu. L'effort de défense représentait 1,82 % du PIB en 2019. Une récession de l'ordre de 10 % portera naturellement cet effort à 2 %, avant même l'échéance de 2025 fixée par la LPM. Si l'économie décroît, les risques stratégiques ne connaissent, eux, aucune décroissance. C'est sur C'est sur ces risques que doit être indexé l'effort de défense, et non sur un PIB qui s'effondre. L'indicateur de 2 % n'est de notre point de vue plus tout à fait adapté. Nous comptons

pour qu'au-delà de 2021 l'effort continue d'être, dans la durée, à la hauteur des enjeux : la force de nos armées et la paix en dépendent. La parole

pendant quelques années, notre pays a cru pouvoir faire bon marché de sa tranquillité. La dynamique s'est récemment inversée, et c'est heureux. Avec le Brexit, et même si des coopérations se poursuivent, l'armée française demeure en effet la seule armée d'envergure au sein de l'Union européenne. La France participe activement à la protection du continent, notamment depuis les pays Baltes. Cette défense nécessite également d'anticiper le développement de menaces, parfois hors de nos frontières. Nos soldats luttent ainsi dans la bande sahélo-saharienne et au Levant contre les groupes armés terroristes, et ce pour la sécurité des populations locale, européenne et française. En plus de ces opérations extérieures, notre armée s'est progressivement vu confier des missions intérieures dans le cadre du plan Vigipirate, mais aussi dans celui de la lutte contre la pandémie. Force est donc de constater que, si notre armée joue pleinement son rôle dans la protection des Français, elle ne se bat pas seulement pour assurer la sécurité de notre nation. Devant l'étendue de la tâche, il est impératif que nous nous assurions que nos soldats disposent des moyens suffisants pour mener à bien leurs missions. Si la pandémie a vocation à prendre progressivement fin, rien ne permet cependant de penser que le niveau d'engagement de l'armée sur d'autres missions est appelé à diminuer à l'avenir. Dans un contexte instable, les Français comme les Européens devront en effet assurer eux-mêmes leur sécurité. Si nos partenaires européens venaient à rester immobiles sur le sujet de la défense, la France aurait encore davantage intérêt à continuer d'entretenir et de renforcer ses capacités militaires. Nous nous félicitons à cet égard que la trajectoire poursuive les objectifs fixés par la LPM. L'actualisation de nos objectifs restera particulièrement importante pour que nous disposions en permanence des moyens d'assurer notre sécurité, dans un contexte toujours changeant. La situation économique constitue une source majeure de préoccupation, car une croissance durablement diminuée mettra en péril le financement de notre force : 2 % d'un PIB amputé par la récession seront-ils suffisants pour affronter les menaces qui pèsent sur nous ? Ces menaces sont évolutives, mais force est de constater que la tendance générale est à la montée des tensions, que ce soit en Méditerranée, en Afrique ou encore en Orient. « L'armée, c'est la nation », disait Napoléon. L'une et l'autre doivent donc se soutenir. Nous regrettons que le plan de relance ne prévoie pas davantage de mesures en faveur du développement de nos capacités militaires. Nous avons pourtant la chance d'avoir en France une industrie de défense de pointe. Le monde nous l'envie, et nous l'envie parfois activement, comme nous l'a montré la récente tentative d'acquisition de la start-up Preligens. Nous avons la possibilité de créer de véritables synergies en investissant pour notre défense, de développer des matériels et des savoir-faire de pointe tout en soutenant l'économie et l'emploi en France. Ne négligeons pas ces opportunités. Nous sommes par ailleurs très attentifs aux conditions de vie de nos soldats, notamment au sort qui sera réservé au Val-de-Grâce. Le logement des militaires en Île-de-France doit être amélioré. Les années à venir seront difficiles à bien des égards. Pour assurer notre tranquillité et celle de nos alliés, nous devrons veiller à continuer d'investir suffisamment pour nos armées.

de l'État », Michelle Gréaume a souligné le déséquilibre entre l'évolution des moyens de notre diplomatie et celle, beaucoup plus rapide, des moyens de défense. La trajectoire de la LPM, en forte augmentation depuis trois ans, dont l'accélération est prévue de façon plus nette encore dans la seconde partie de sa mise fait en quelque sorte de nos armées notre vitrine diplomatique. Est-ce bien là le sens que nous devrions donner à l'action extérieure de la France ? Notre budget militaire, avec une augmentation de 4,5 % cette année, atteint 39,2 milliards d'euros. On peut, comme vous le ferez, madame la ministre, se féliciter de cette augmentation programmée et respectée. On peut aligner les chiffres de la livraison promise et effective de nouveaux équipements : Griffon, Jaguar, fusils d'assaut, nouveaux avions MRTT (), hélicoptères, frégates ces chiffres contiennent une part de remise à niveau nécessaire de nos capacités opérationnelles et de nos équipements, mais aussi du traitement et de la condition de nos militaires et de leurs familles : je pense au plan Famille, à l'hébergement, à l'augmentation des soldes, aux petits équipements.

Je veux insister sur un point : l'autosatisfaction sur des dépenses en augmentation ne suffit pas à dire, dans ce monde bouleversé et mouvant, si nous sommes sur la bonne trajectoire en matière de défense, quand tant d'incertitudes et d'évolutions géostratégiques nous interrogent.

Ce que nous construisons d'abord et surtout, c'est une armée massivement tournée vers la présence et les opérations extérieures. Ainsi, 13 000 de nos militaires sont déployés sur le territoire national, quand 5 100 le sont au Sahel dans l'opération Barkhane. Il y en a également 3 750 dans nos bases militaires au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Gabon, à Djibouti et aux Émirats arabes unis, 600 dans l'opération Chammal en Irak et Syrie, 4 500 en mission maritime sur les mers du monde et 400 auprès de l'OTAN. La structure de déploiement vers laquelle nous ne cessons d'évoluer est donc claire et elle mériterait pour le moins un débat stratégique. J'espère par exemple que nous pourrons débattre de la poursuite, ou non, de l'opération Barkhane.

L'« autonomie stratégique européenne », nous répète le Président de la République. Or c'est exactement le contraire de ce que vient de déclarer la ministre allemande de la défense, qui parle d'en finir avec « l'illusion de l'autonomie stratégique » et pour qui l'OTAN reste l'unique boussole stratégique.

ou plutôt de la relance de programmes tournés vers l'exportation et la vente d'armes, guidés par l'engrenage d'une hypersophistication technologique, génératrice de surarmement

stratégique, ainsi qu'à la reconstruction d'une filière nationale de production de munitions de petit calibre. Le paradoxe est que nous n'en avons plus, alors que Thales aide l'Australie à s'en construire une Enfin, j'en viens à l'avenir de notre dissuasion nucléaire, dans laquelle nous investissons cette année 5 milliards d'euros, sans compter le coût de lancement des études sur un nouveau porte-avions. Cela mérite un débat approfondi et sans tabou, au moment où s'approchent de nouvelles ruptures technologiques et où la fin du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, dénoncé par Donald Trump, risque de conduire à une nouvelle escalade extrêmement inquiétante. Vous l'aurez compris, madame la ministre, c'est plus d'une revue d'intérêt stratégique de nos priorités budgétaires que d'une litanie de crédits à la hausse que nous estimons avoir besoin. La relance tous azimuts

Cette opération a été la contribution des armées contre la propagation du virus. Centrée sur l'aide et le soutien aux populations, ainsi que sur l'appui aux services publics pour faire face à cette épidémie en métropole et en outre-mer, elle a apporté un soutien déterminant dans les domaines de la santé, de la logistique et de la protection. Elle a permis le transfert de 146 patients pour décongestionner les services de réanimation de l'est de la France, ainsi qu'une meilleure répartition des personnels soignants.

Après des décennies de déflation, la LPM entend accorder des moyens aux armées, afin de remédier aux carences du passé et de permettre une remontée en puissance, tout en préparant l'avenir d'une défense nationale adaptée aux défis et conflits du XXI siècle.

Vous aviez le choix entre le déshonneur et la guerre ; vous avez choisi le déshonneur, et vous aurez la guerre. » Il est donc extrêmement important- certes, on sait que c'est difficile -de définir une politique lorsque des conflits

Je pense par exemple à la décision du Président de la République d'envoyer dans le cadre l'opération Barkhane, en début d'année, 600 soldats supplémentaires en renfort dans la zone dite des trois frontières, au Sahel, en plus des appuis aériens. Le budget pour 2021 de la mission « Défense » respecte les engagements pris dans le cadre de la LPM 2019-2025. Alors que le risque de conflit dans le monde s'accroît et que la France connaît une crise économique liée à la crise sanitaire dont on ne connaît pas encore toute l'ampleur, il était impératif de ne pas raboter le budget des armées et d'en refaire, comme autrefois, une variable d'ajustement. Face à un monde de plus en plus instable et dangereux, renoncer aux moyens de sa puissance et de sa protection serait de la folie. Répondant à ces besoins importants et croissants, et restant fidèle à la trajectoire tracée par la LPM, le projet de budget que nous examinons est au rendez-vous des engagements pris. Il prévoit en effet une augmentation de 4,5 % par rapport à 2020, avec 1,7 milliard d'euros des moyens accordés à la défense, hors contribution au compte d'affectation spéciale « Pensions Sur le plan capacitaire, nous nous félicitons et saluons la livraison de nombreux équipements, ainsi que les différentes commandes prévues en 2021. Je pense par exemple aux systèmes de drones tactiques SDT, aux engins blindés de reconnaissance ou encore aux avions de transport et de ravitaillement A330 MRTT Phénix. Il s'agit ici de signes visibles et concrets de la remontée en puissance des armées. Cette arrivée de matériels témoigne des efforts et des progrès accomplis en termes d'innovation. Vous l'aurez compris, madame la ministre, nous sommes plutôt satisfaits à la lecture de ce budget. Cependant, je souhaite appeler votre attention sur quelques points de vigilance. Le premier de ces points, et non des moindres- il a été évoqué -, est la question de l'actualisation de la loi de programmation militaire.

À l'occasion de l'examen des crédits de la mission « Défense », pouvez-vous nous en dire plus ? Nous nous interrogeons également sur le prochain porte-avions de nouvelle génération, qui aura vocation à remplacer le à l'horizon 2038. Les arbitrages sur ce dossier seront-ils rendus prochainement ? Cette année encore, le projet de loi de finances initiale est grevé par le surcoût généré par les OPEX et les missions intérieures (Missint). En 2020, ce surcoût intègre notamment le renforcement des effectifs de l'opération Barkhane,

Je souhaite également revenir sur la fidélisation de nos forces. Les crédits de personnels sont en hausse de 179 millions d'euros dans ce projet de loi de finances, ce qui représente une augmentation de 1,5 %. L'année 2021 sera en effet la première année de la mise en oeuvre de la nouvelle politique de rémunération des militaires. Le plan Famille, lancé voilà trois ans, est essentiel à cette démarche de fidélisation. En 2021, il se traduira par la poursuite des efforts en matière de construction d'hébergement, de crèches et de logements, en métropole comme en outre-mer, d'amélioration des conditions de vie en garnison, d'action sociale et d'accompagnement des conjoints à l'emploi ou à la mobilité. Si certaines de ses mesures sont perçues très positivement par les militaires, des avis plus contrastés ont été exprimés sur la situation du logement et les conditions d'hébergement dans les enceintes militaires. Dans son rapport spécial fait au nom de la commission des finances, Dominique de Legge, dont je salue ici le travail, ainsi que celui de tous les rapporteurs pour avis, estime même que tout cet effort de fidélisation pourrait être compromis par le retard pris en matière d'infrastructures et de logement. La question des pensions de retraite militaires fera également l'objet d'un suivi très scrupuleux de la part de notre commission. Enfin, nous ne pouvons que constater que la défense est la « grande oubliée » du plan de relance. Elle n'est concernée qu'au titre de l'accélération des commandes d'aéronefs, à hauteur de 600 millions d'euros. Le plan de relance vise à soutenir les secteurs qui souffrent et à provoquer un effet levier. Or cet effet est généralement particulièrement dynamique dans l'industrie de la défense. Dans ce secteur d'activité, l'efficacité de l'investissement public en matière d'emploi est bien supérieure à ce qu'elle est dans tous les autres. Madame la ministre, le groupe UC votera les crédits de la mission « Défense » et sera tout à fait attentif à l'évolution des points soulevés dans cette intervention. La

avec 39,2 milliards d'euros, en hausse de 4,5 %, le projet de budget des armées pour 2021 apparaît toujours comme une priorité nationale. La loi de programmation militaire 2019-2025 est respectée, ce dont je ne peux que me féliciter. féliciter. À y regarder de plus près toutefois, c'est l'arrêt des usines d'armement pendant le confinement qui a facialement préservé l'exercice 2021, puisque cela a conduit le ministère à ne pas dépenser 1,1 milliard d'euros de crédits. Ces crédits non consommés ont permis de couvrir les dépenses nouvelles de 2020, notamment les surcoûts des opérations extérieures. Ces derniers devraient atteindre un record inégalé, avec 1,6 milliard d'euros à la fin de l'année 2020, soit 500 millions d'euros de plus que prévu, en raison du renforcement de l'opération Barkhane, de l'opération de secours menée au Liban, mais également du soutien à la lutte contre le covid. Il faut y ajouter les surcoûts liés aux missions intérieures, avec la montée en puissance de l'opération Sentinelle et ses 7 000 soldats mobilisés.

Cette opération risque de laisser un surcoût pour l'armée évalué à 1 milliard d'euros. Le produit de la vente de ces Rafale est estimé à 400 millions d'euros. Si la possibilité d'une rétrocession de ces produits un compte d'affectation spéciale a été évoquée, les recettes de vente seront inscrites au budget général de l'État, et non au budget du ministère des armées. Certes, madame la ministre, il vous revient de négocier la rétrocession de cette vente, mais cette négociation entre votre ministère et Bercy est loin d'être garantie. Enfin, l'autre conséquence immédiate est l'affaiblissement de nos capacités opérationnelles d'ici à 2025 retirer 12 Rafale sur 102, c'est diminuer la flotte de plus de 10 %. Madame la ministre, avez-vous signé le bon de commande pour les Rafale au profit de nos armées ?

millions d'euros et inclut la réparation de la Perle et la prolongation du Rubis. Rapporté au budget global de la défense, ce coût représente un choc financier majeur.

ainsi qu'un plan de rattrapage capacitaire, la situation est très préoccupante : fragilisation des chaînes de production, difficultés avec les banques, fonte des marchés à l'export,

alors que la LPM mise sur son développement. L'autonomie stratégique européenne nécessite de partager une vision commune des menaces, mais aussi d'avoir la volonté de renforcer l'indépendance et la capacité d'innovation des industries européennes du secteur. Or le Fonds européen de défense est reconduit avec un budget amputé de moitié. Est-ce un bon signe à adresser à nos partenaires, en particulier allemands ? Je ne le crois pas. Comment, dans un tel cadre, rester compétitifs en matière de recherche et d'innovation technologique, alors que l'Europe est confrontée à un environnement de plus en plus compétitif ? La culture commune en matière de défense est à construire. Il est nécessaire que toutes les initiatives nationales

Cette coopération européenne doit aussi se traduire dans les faits. Au mois de février dernier, la France et l'Allemagne ont lancé la première phase du programme de

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je salue à mon tour la mémoire de nos militaires disparus et rends hommage à l'engagement de tous ceux qui participent à la défense de notre pays et oeuvrent pour la paix et la sécurité, en France et à l'étranger, ainsi qu'à leur famille. N'oublions jamais en effet que les proches d'un militaire représentent le soutien indispensable et l'ancrage qui participe aussi à la réussite de leur mission. Madame la ministre, vous nous présentez un budget de la défense pour 2021 conforme à vos engagements et à la trajectoire de la LPM. Nous observons avec satisfaction que les crédits de paiement s'élèvent à 39,2 milliards d'euros, soit une augmentation de 1,6 milliard d'euros, dont une grande part sera consacrée au programme 146. Ce fléchage vers le renouvellement des matériels est à souligner du fait de la très grande attrition et de l'obsolescence des matériels utilisés sur les théâtres d'OPEX. Il faut une politique de maintien capable de mieux anticiper les besoins des hommes sur le terrain. Il y va du principe même de notre capacité opérationnelle. Des efforts ont été réalisés en amont avec les industriels, et nous nous en félicitons. Néanmoins, la question se pose encore plus avec les conséquences de la covid, qui n'ont pas épargné l'industrie française de défense, grands groupes ou PME, en France et à l'étranger, avec un lourd impact sur les trésoreries et les capacités de production. de l'armement (DGA) en direction des 1 000 PME sous-traitantes des fournisseurs sont bienvenus, mais restent insuffisants en comparaison des autres pays, dont les usines ont poursuivi leur activité. Nous regrettons que le plan de relance ne concerne la défense qu'au titre de l'accélération de commande d'aéronefs, et pour 600 millions d'euros. À cela s'ajoutent les très grandes difficultés pour les sociétés françaises à trouver des soutiens financiers, les banques restant trop frileuses vis-à-vis du secteur de la défense. C'est ubuesque. À titre de comparaison, les Britanniques ont annoncé qu'ils consacreront à leur défense près de 27 milliards d'euros sur les quatre prochaines années, ce qui en fait le deuxième contributeur budgétaire au sein de l'OTAN, après les États-Unis. Cette décision, qui n'est pas seulement liée au Brexit, entraînera la création de 10 000 emplois et de nouvelles capacités, quand nous supprimons des postes militaires dans nos ambassades. Pourtant, avec la dégradation de l'environnement sécuritaire, jamais nous n'en avons eu autant besoin. Sur le volet capacitaire toujours, comment imaginer que nos capacités resteront inchangées à la suite du prélèvement des 18 avions Rafale sur la flotte de l'armée de l'air ? C'est l'incarnation de la politique du « en même temps » : d'un côté, vous augmentez les crédits des programmes 146 et 144 ; de l'autre, vous amputez l'armée de l'air de 25 %. Comment obtenir la garantie que le produit de cessions des Rafale à la Grèce reviendra au budget des armées, alors même qu'il ne bénéficie plus de la solidarité interministérielle pour le financement des OPEX ? Il y avait l'option d'un compte d'affectation spéciale, mais ce serait un retour en arrière en termes de « sincérisation » budgétaire, car c'est un retour à la logique du financement par recette exceptionnelle, comme sous le précédent quinquennat. En outre, nous devons reconnaître- hélas ! -que notre soutien matériel à la Grèce est lié à une incapacité politique et stratégique de l'Alliance et de l'Union européenne vis-à-vis de la Turquie. En tant que vice-présidente de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, très attachée aux valeurs de l'Alliance, je ne peux que regretter la faiblesse des réactions de cette organisation, de l'Union européenne et de leurs États membres face à des agressions caractérisées envers un autre État membre, Chypre, et envers des pays partageant les valeurs otaniennes, comme l'Arménie. Dans cette affaire, la France subit une double peine : du point de vue diplomatique et du point de vue de son outil militaire. outil militaire. La politique de fidélisation des armées, enjeu majeur pour leur avenir, constitue un autre sujet primordial. Recruter, c'est bien ; préserver et conserver les effectifs, c'est mieux. Pour cela, la mise en place d'une véritable politique dédiée au quotidien des familles prenant en compte la spécificité de l'état militaire est cruciale. Nous saluons les 95,5 millions d'euros pour 2021 pour le renouvellement du parc locatif et l'augmentation des places d'hébergement, notamment dans les zones tendues. Sur ce point, madame la ministre, pourriez-vous nous dire où en sont les discussions avec la maire de Paris ? Le Val-de-Grâce, contre la fermeture duquel je m'étais beaucoup élevée, sera cédé en 2024. Pour quoi, à qui et pour combien ? Pourquoi ne pas l'avoir réhabilité pour les acteurs de la défense ? N'oublions pas non plus que les infrastructures dédiées à l'hébergement des militaires doivent répondre à des critères de sécurité, les militaires étant eux-mêmes des cibles.

Monsieur le président, monsieur le président de la commission, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs,

en est le socle. N'oublions pas que le président Giscard d'Estaing avait un lien particulier avec nos armées. Il s'était engagé à dix-huit ans pour la libération de Paris, puis dans la Première armée.

Chacun le sait, c'était un ancien élève de l'École polytechnique. Lorsqu'il accéda, en 1974, à la présidence de la République, il engagea une profonde modernisation de nos forces armées. Au cours de son septennat, une loi de programmation militaire fut adoptée.

dans cette loi de programmation 1977-1982 qu'a été prise la décision de lancer le programme des sous-marins nucléaires d'attaque Rubis.

un signe tout à fait marquant de la continuité des actions et des décisions qui sont prises pour la France. C'est avec une grande fierté que je vous présente le projet de budget pour 2021 de la mission « Défense », qui, pour la troisième année consécutive, respecte à la lettre les engagements et la trajectoire financière de la loi de programmation militaire. Ce budget est la marque du respect de l'engagement fort du Président de la République de porter l'effort national de défense à 2 % de la richesse nationale d'ici à 2025. Cet objectif n'est pas seulement symbolique. Il poursuit et consolide la remontée en puissance de nos armées, engagée par la loi de programmation militaire. vous l'avez noté dans vos interventions, l'objectif de 2 % du PIB pourrait être atteint dès 2020 en raison des effets de la crise sanitaire sur notre économie. Pour autant, c'est une conséquence purement arithmétique de la crise. Cela signifie-t-il que nous avons suffisamment modernisé nos armées et qu'elles sont désormais mieux équipées ? sûr que non ! L'effort doit se poursuivre, et il se poursuit. Vous avez soulevé dans vos interventions la question de l'actualisation de la loi de programmation militaire. Cette dernière doit avoir lieu au plus tard en 2021. Le travail de préparation est en cours sur le fondement d'une mise à jour de notre analyse du contexte géostratégique nous permettant d'identifier les ajustements envisageables pour répondre à l'évolution de la menace et des risques. Conformément à la loi de programmation militaire, les crédits pour le ministère des armées s'élèveront à 39,2 milliards d'euros en 2021, soit 7 milliards de plus qu'en 2017.

Dans le contexte actuel, ce budget 2021 est une contribution essentielle à la relance économique de notre pays. Si l'on raisonne plus globalement, sur la première partie de la LPM, 110 milliards d'euros auront été injectés dans l'économie pour les équipements, les infrastructures et le maintien en condition opérationnelle. C'est donc l'équivalent en cinq ans d'un plan de relance pour les seules questions de défense. ailleurs un plan de relance qui s'adapte : dès le mois de juin dernier, pour venir en aide au secteur aéronautique durement touché par la crise sanitaire, nous avons accéléré certaines commandes prévues au cours de la LPM, pour un montant de 600 millions d'euros.

précise que, si le contrat aboutit, le produit de la vente des Rafale d'occasion reviendra au budget du ministère des armées. Nous avons eu toutes les assurances du ministère de l'économie et des finances à ce sujet. Naturellement, nous nous organisons pour que la vente des avions issus de nos forces à l'armée de l'air grecque

La loi de programmation militaire fixe une ambition capacitaire pour l'armée de l'air et de l'espace, comme pour les autres armées. Cette ambition sera respectée.

complétée par celle de 12 Rafale neufs par l'armée de l'air et de l'espace française pour compenser les prélèvements réalisés au profit de la Grèce,

Pour en revenir au budget, le ministère des armées sera en 2021 une véritable fabrique de l'emploi : il sera le premier recruteur de l'État, avec près de 27 000 recrutements, soit 300 de plus que l'année précédente. L'effort en termes d'apprentissage sera poursuivi. Nous recruterons des jeunes venus de tous les territoires de notre pays et de tous les niveaux de formation. Nous Nous poursuivrons également l'effort engagé dans les domaines du renseignement, du cyber et du numérique. J'en viens au détail du contenu du budget et je vous propose de l'examiner en reprenant les quatre axes de la loi de programmation militaire.

Ceux qui ont eu la chance de se rendre en opération sur le terrain ont pu constater qu'en 2020, conformément à l'objectif fixé, 100 % de nos soldats déployés en OPEX en sont équipés. Troisièmement, nous modernisons la solde. Avec 38 millions d'euros dans le budget 021, nous amorçons la nouvelle politique de rémunération des militaires, avec un dispositif renforcé d'indemnisation de la mobilité géographique.

J'ai décidé cette année d'augmenter le budget de ce service de 160 millions d'euros d'ici à la fin de la LPM. Cette décision s'inscrit dans la dynamique de l'effort entamé depuis 2017, lorsque nous avons mis fin- enfin ! -à la déflation des effectifs du service de santé des armées. Nous avons également pris plusieurs mesures de revalorisation salariale au profit des praticiens et du personnel paramédical, à hauteur de 31 millions d'euros entre 2017 et 2020. Une question a été posée sur les mesures de protection que nous prenons à l'égard de nos militaires lorsque ceux-ci partent en opération ou en mission.

Il me semble que nous avons progressivement trouvé les méthodes qui permettent de préserver la santé de nos militaires et de leurs familles, mais aussi des populations au contact desquelles ils peuvent être amenés à évoluer.

Nous consoliderons également les commandes de 21 hélicoptères interarmées légers et 120 véhicules blindés légers. Pour la marine, 2021 verra notamment la livraison de 3 avions de patrouille Atlantique 2 rénovés et d'une nouvelle frégate multimissions. Nous engagerons les commandes d'une nouvelle frégate de défense et d'intervention ainsi que de 8 hélicoptères légers. Comme la question du porte-avions de nouvelle génération a été abordée, je tiens à vous rassurer. Nous avons travaillé vite, nous ne sommes absolument pas en retard. Nous avons réalisé au cours des deux dernières années des études

Enfin, l'armée de l'air et de l'espace réceptionnera en 2021 3 avions ravitailleurs MRTT Phénix, 14 avions de chasse mirage M2000D rénovés et un avion de transport A400M supplémentaire. supplémentaire. Les commandes concerneront le lancement du démonstrateur du système de combat aérien du futur. Le troisième chapitre de la LPM concerne la consolidation de notre autonomie stratégique. Ce budget 2021 y contribuera, notamment avec 5 milliards d'euros pour poursuivre le renouvellement des deux composantes de la dissuasion française. Le ministère des armées poursuivra son effort en faveur de la stratégie spatiale, en lui allouant 624 millions d'euros. J'ai souhaité faire de l'espace une priorité de la loi de programmation militaire et ai donc proposé au Président de la République une stratégie spatiale de défense à la hauteur des défis qui se présentent à nous. Nous y consacrons des moyens considérables : 4,5 milliards d'euros pour la période 2019-2025. En 2021, le secteur spatial verra notamment la livraison d'un satellite MUSIS/CSO. Je tiens à cette occasion à remercier

J'en viens enfin au dernier chapitre de la LPM, la préparation du futur : 2021 sera l'année de la commande du démonstrateur du système de combat aérien du futur que nous construisons avec les Allemands et les Espagnols. Celui-ci devrait prendre son envol en 2026, pour être opérationnel à l'horizon 2040.

Pour répondre à une question qui a été posée, l'Espagne est un partenaire important, d'ores et déjà intégré aux travaux d'architecture et de recherche et développement, qui avaient été initialement lancés dans un cadre franco-allemand. Pour la phase du démonstrateur, qui devrait être lancé d'ici à la mi-2021, l'Espagne sera un contributeur majeur, aux côtés de la France et de l'Allemagne. La préparation du futur passe aussi par l'innovation : en 2021, nous consacrerons près de 900 millions d'euros pour concevoir les technologies de demain et nous serons donc en bon chemin vers le milliard d'euros annuel qui sera atteint en 2022. L'année 2021 sera également celle de la mise en oeuvre du nouveau Fonds Innovation défense, qui viendra compléter les mécanismes existants de soutien aux PME, tels que le dispositif Rapid. Ce nouveau fonds sera doté de 200 millions d'euros pour soutenir le développement des technologies duales et transversales, par le financement en fonds propres d'entreprises innovantes.

J'ai demandé au délégué général pour l'armement d'examiner avec les organisations professionnelles des industries de défense, les services de Bercy et les représentants de la profession bancaire l'existence de clauses ou de pratiques

voie le jour. Il sera doté de 7 milliards d'euros constants pour la période 2021-2027. C'est la première fois que des financements européens seront affectés à la recherche et au développement dans le secteur de la défense. Notre devoir Notre devoir à tous est de mettre en oeuvre la loi de programmation militaire, de veiller à son exécution, dans chaque régiment et chaque unité, en métropole comme en outre-mer.

Défense », par des contributions internationales et redéploiements internes, pour un montant total inférieur à 60 millions d'euros et, enfin, par des ouvertures de crédits en loi de finances rectificative, pour 200 millions d'euros. Il faut conclure, madame la ministre. Dans le contexte de la crise sanitaire, j'ai décidé

marque la poursuite de notre mission de protection des Français et de soutien à nos entreprises, nos emplois et nos territoires. Nous allons

On pense forcément à l'élément de réanimation installé à Mulhouse, qui a permis d'accueillir une quarantaine de patients, et de soulager ainsi l'hôpital public. Il serait toutefois injuste de ne pas rappeler le triplement des places en réanimation dans les hôpitaux d'instruction des armées, la mise à disposition de matériel et d'unités de réanimation d'urgence, le transfert organisé de malades ou encore la mobilisation des médecins, d'une partie des élèves et des réservistes du service. On perçoit d'autant mieux les manques qui affligent le service de santé des armées. Comment espérer une pleine mobilisation auprès des malades civils tout en maintenant la protection des militaires en opération extérieure

sont pris en étau entre une distanciation sociale incompatible avec la vie en garnison et la décision gouvernementale de maintenir la quasi-totalité des opérations militaires. Il faut donc un service de santé des armées suffisamment doté pour fonctionner. Or ce n'est clairement pas le cas, malgré l'engagement d'augmenter les effectifs inscrit dans la loi de programmation Il manque aujourd'hui 100 médecins dans le service, alors que son déploiement n'a jamais été aussi important. Après avoir perdu près de 10 % de ses effectifs entre 2013 et 2019, le taux de projection des équipes médicales est de 106 et de 200 % pour les équipes chirurgicales ; et encore, il faut remercier les réservistes, qui assurent environ 15 % du contrat opérationnel.

à 2025. Concernant les praticiens du service de santé des armées, vous avez raison, nous n'arrivons pas à pourvoir l'ensemble des postes.

du matériel de vie en campagne, des rations de combat, bref de tout ce qui détermine les conditions d'exercice du métier des armes de nos soldats. C'est pourquoi le programme 178 voit les dépenses de petit équipement progresser de 95 millions d'euros en 2021.

à l'occasion de cette séance budgétaire, il convient, comme les années précédentes, de rappeler tout d'abord que nos forces de l'ordre connaissent depuis quelques années une tension permanente

Des voitures radars à conduite externalisée seront déployées dans les régions françaises. Les recettes sont estimées à 2 milliards d'euros pour les amendes. À ce sujet, il faut reconnaître que le compte d'affectation spéciale devient de plus en plus opaque et qu'il se doit d'être rapidement réformé et révisé. Il constitue un problème de plus en plus prégnant pour l'ensemble des élus.

Auparavant, comme Jean-Pierre Vogel en a l'habitude, je rends hommage à l'ensemble des sapeurs-pompiers, des pilotes, des formations militaires de la sécurité civile et des associations agréées, qui s'investissent sans compter dans la lutte contre les crises qui touchent notre pays, en particulier la crise sanitaire actuelle. Face à ces crises, il pourrait à première vue sembler paradoxal que les crédits du programme 161, « Sécurité civile », soient stables en 2021. cette stabilité n'est qu'apparente. En effet, une part importante des crédits du programme 161, « Sécurité civile » a été transférée vers la mission « Plan de relance », pour un total d'environ 37,5 millions d'euros. Ce procédé, qui a également été appliqué pour la police et la gendarmerie, laisse songeur. Une bonne partie de ces crédits transférés ne recouvrent pas des mesures de relance. Il s'agit en effet de dépenses ordinaires, qui financent par exemple le maintien en condition opérationnelle (MCO) de nos avions. je relève aussi que ce plan de relance financera des projets d'envergure pour la sécurité civile. Je pense notamment aux 50 millions d'euros qui iront au « 112 inversé pour prendre la suite du volet mobile du système d'alerte et d'information des populations (SAIP). À cet égard, Jean-Pierre Vogel salue le choix de la technologie de. Il l'avait

Cela étant, ces crédits portés par le plan de relance nuisent à la lisibilité de l'effort financier de l'État en faveur de la sécurité civile, effort qui est déjà très éclaté. Au total, ce sont dix programmes, répartis dans huit missions et pilotés par six ministères différents, qui concourent au financement de notre politique de sécurité civile, à hauteur de 1,2 milliard d'euros pour 2021. Comble de cette dispersion des crédits, la contribution du programme 161, « Sécurité civile », sera minoritaire, puisqu'il représente 43 % de l'effort total, contre la moitié ces dernières années. Le programme 161 ne recouvre aussi qu'une infime partie des moyens des Ces derniers totalisent 5 milliards d'euros de dépenses en 2019. La croissance de leurs charges n'est toutefois pas toujours de leur fait, comme l'illustre le cas de la revalorisation de la prime de feu, qui représente un surcoût global de 80 millions d'euros. Il est satisfaisant que le Gouvernement ait tenu ses engagements sur ce point, avec la suppression de la surcotisation patronale versée à la Caisse Il s'agit toutefois d'une compensation partielle, et non d'une économie nouvelle, comme cela a pu être présenté à tort. Ainsi, malgré cette mesure, le surcoût se situera toujours entre 30 millions d'euros et 40 millions d'euros pour les SDIS.

Pour cela, la mise en place du 112 comme numéro unique pour les appels d'urgence doit être privilégiée. Il faut aussi encourager la création des plateformes communes de traitement des appels, comme s'y était engagé le Président de la République, il y a trois ans. Enfin, un intérêt particulier doit être porté à la flotte de la sécurité civile. Son vieillissement a de quoi nous préoccuper, tant elle se révèle cruciale en ces temps de crise. Ce projet devrait certes y remédier en partie, avec la poursuite de la commande des nouveaux avions Dash et la livraison de deux d'entre eux l'an prochain. prochain. Jean-Pierre Vogel a maintes fois souligné combien le choix de ce modèle d'avion était pertinent : les récents retours d'expériences tendent à le confirmer. Il est également satisfaisant que la France puisse bénéficier d'un cofinancement de l'Union européenne pour acquérir deux nouveaux avions Canadair, et peut-être même un hélicoptère bombardier d'eau. Vous en conviendrez, madame la ministre, ces financements extrabudgétaires ne doivent cependant pas nous dispenser de maintenir un niveau suffisant de crédits pour la modernisation et le renouvellement de notre flotte.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette année, le père Noël est passé plusieurs fois pour les gendarmes Si nous additionnons la loi de finances rectificative, ce projet de loi de finances et le plan de relance, la gendarmerie va pouvoir acquérir au total près de 6 000 véhicules, dont dix hélicoptères H160. L'immobilier constitue sans doute une préoccupation plus importante encore pour les gendarmes. Les crédits du projet de loi de finances, qui n'évoluent quasiment pas, devraient toutefois être complétés par ceux du plan de relance, à hauteur de 440 millions d'euros.

Les projets doivent en principe être livrés dans les deux ans, trois au maximum, ce qui sera un peu court pour certaines opérations complexes. Des dérogations seront-elles possibles ?

Or le futur projet de loi sur la sécurité intérieure, qui pourrait comporter une telle programmation, n'est annoncé que pour 2022. Deuxièmement, la réserve opérationnelle est devenue essentielle à la gendarmerie nationale, que ce soit durant la période estivale dans les zones d'affluence saisonnière ou lors de certains grands événements nationaux, mais aussi, par exemple, dans la lutte contre l'immigration illégale. Il existe

De l'autre, les crédits stagnent, ce qui retarde l'emploi des réservistes déjà recrutés. Dès lors, il est impératif d'assurer une remontée en puissance des crédits de la réserve opérationnelle et d'offrir à celle-ci une visibilité à moyen et long termes.

madame la ministre, mes chers collègues, certes, l'augmentation des effectifs et des crédits d'investissement de la gendarmerie pour 2021 est une satisfaction, mais nous restons extrêmement inquiets au regard d'une certaine absence de visibilité pour les prochaines années.

Cette déclaration soulève des interrogations, voire suscite une certaine inquiétude. Il est en effet toujours nécessaire d'observer la plus grande prudence sur ce genre de réformes, même si, en l'occurrence,

de la gendarmerie a déjà évolué au cours des dernières années, notamment dans le cadre de la révision générale des politiques publiques (RGPP), avec la fermeture de nombreuses casernes. Or ces évolutions ont parfois remis en cause une adaptation fine aux réalités de la délinquance, qu'un travail de plusieurs années avait permis d'obtenir. C'est notamment le cas lorsque des brigades de gendarmerie ont laissé place à la police dans des zones périurbaines. En tout état de cause, la consultation préalable des élus locaux concernés, évoquée par le Livre blanc, devra être organisée de manière efficace, afin de bénéficier de leur connaissance des besoins de la population.

Les crédits de la réserve constituent trop souvent une variable d'ajustement. Chaque année, la mise en réserve de 4 % des crédits hors titre 2 et le surgel ministériel de 1 perturbent gravement l'exécution budgétaire, puisque près des deux tiers des dépenses de la gendarmerie sont obligatoires. M. le ministre,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je vous prie de bien vouloir excuser Henri Leroy, que je tenterai de remplacer au mieux pour présenter ses conclusions. Une fois n'est pas coutume, la semaine dernière, la commission des lois a donné un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission « Sécurités » inscrits au projet de loi de finances pour 2021. Nous devons reconnaître que ce projet de loi rompt avec les orientations budgétaires des dernières années, qui ont consisté à mettre l'accent sur le renforcement des effectifs, au détriment de l'amélioration des conditions de travail de nos forces de sécurité. Pour la première fois, en effet, le budget apporte une réponse à la hauteur des revendications et des besoins de nos policiers et gendarmes. Cette évolution positive n'est pas liée à la mission « Sécurités » en elle-même, laquelle est, une nouvelle fois, assez décevante. Hors programme « Sécurité civile », les crédits de paiement de la mission connaissent en effet une hausse de seulement 1,2 1,2 % par rapport à 2020, bien plus faible que les années précédentes. Nous avons cependant pris acte de l'abondement important dont les forces de sécurité devraient bénéficier au titre du plan de relance, même si nous regrettons le manque de lisibilité sur le contenu exact de ce plan. Selon les informations dont nous disposons, ces moyens supplémentaires permettront de faire progresser les dépenses de fonctionnement et d'investissement de plus de 11 % dans la police et de 12 % dans la gendarmerie par rapport à l'exercice 2020. Il s'agit d'évolutions sans précédent depuis plusieurs années. Ces augmentations permettront, nous l'espérons, de combler les retards pris dans l'équipement des forces de sécurité intérieure. Philippe Dominati en a donné le détail. Il s'agira notamment de réaliser un effort important sur les renouvellements de véhicules, sur les équipements individuels et sur la rénovation du parc immobilier. Comme la commission des finances, la commission des lois s'est félicitée de ces évolutions. Elle a toutefois souhaité mettre en avant deux points qui doivent appeler l'attention. Le premier point porte sur l'impact du plan de recrutements engagé par le Gouvernement. Nous ne remettons pas en cause le besoin d'effectifs complémentaires, mais nous contestons la méthode. Nous le savons, les recrutements massifs des dernières années ont engorgé les systèmes de formation et se sont traduits par un épuisement des viviers de recrutement, avec des conséquences dommageables sur le niveau de nos jeunes forces de l'ordre. Madame la ministre, d'autres voies doivent être approfondies pour alléger la tâche des forces de l'ordre : nous pensons non seulement à l'approfondissement des réformes structurelles, mais également à une mobilisation plus importante des réserves. Le second point concerne l'avenir. Le projet de loi de finances pour 2021 constitue, à notre sens, un bon budget pour les forces de sécurité. C'est pourquoi nous avons décidé d'y donner un avis favorable. Cependant, nous devons rester attentifs à ce que cet effort s'inscrive dans la durée. Nos forces de sécurité ont en effet besoin de perspectives pour remettre à niveau leurs équipements et se moderniser. Il s'agit non seulement d'une reconnaissance de leur engagement, mais également d'une condition pour assurer la sécurité de nos concitoyens.

qui bénéficieront aux moyens nationaux de la sécurité civile augmentent. C'est la raison pour laquelle elle a émis un avis favorable à leur adoption. Au-delà de cet avis favorable, je formulerai trois remarques sur les crédits du programme 161, « Sécurité civile En tant que sénatrice récemment élue, je me confronte pour la première fois à l'exercice budgétaire. Force est de constater que ce premier contact est étourdissant Devant un programme explicitement intitulé « Sécurité civile », nous pourrions naïvement penser qu'il regroupe l'ensemble des crédits destinés aux moyens nationaux de la sécurité civile. Cela est faux, puisque ce programme en représente à peine 40 il doit être lu à la lueur des huit autres programmes qui alimentent la politique transversale « Sécurité civile », à la lueur de la mission « Plan de relance », ainsi qu'à la lueur des crédits en lien avec la sécurité civile essaimés à l'occasion des différentes lois de finances rectificatives.

ma deuxième remarque, le budget que l'État consacre à la sécurité civile doit être rapproché du budget global des SDIS, qui s'élevait, en 2019, à plus de 5 milliards d'euros, presque exclusivement à la charge des collectivités, au premier rang desquelles se trouvent La qualité de la politique nationale de sécurité civile est donc largement tributaire des moyens dont disposent nos SDIS et de ceux des collectivités territoriales, les départements en tête. Il se trouve que la santé financière de ces derniers va nécessairement pâtir de l'actuelle crise sanitaire. Face à ces difficultés à venir, il est primordial de rationaliser les dépenses de nos SDIS. À ce titre, la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises qui permettrait de mutualiser certaines dépenses entre SDIS. Je salue cette initiative, mais constate que de nombreux efforts de mutualisation ont déjà été mis en oeuvre entre nos SDIS. Je crains donc que les économies restant à réaliser soient décevantes. En revanche, j'appelle la DGSCGC à une très grande vigilance dans l'élaboration des référentiels techniques qu'elle pourrait être amenée à mettre en oeuvre dans les mois à venir. Je souhaite que les changements de normes induisant le remplacement du matériel des SDIS soient réduits au strict nécessaire, afin d'éviter les surcoûts de nouvelles acquisitions. Enfin, ma troisième remarque porte sur la philosophie avec laquelle il faut analyser le coût de la sécurité civile. Devant la raréfaction à venir des deniers publics tant pour l'État

qu'elle permet de réaliser, à tout niveau, afin de considérer ce coût pour ce qu'il est : un investissement et non une perte sèche. Une prise de conscience de ce gain réel est nécessaire, pour que tous les acteurs de la sécurité civile bénéficient de moyens adéquats afin d'assurer leurs missions d'intérêt général. Mes Mes chers collègues, je vous rappelle que le temps de parole attribué à chaque groupe pour chaque unité de discussion comprend le temps d'intervention générale et celui de l'explication de vote. Par ailleurs, le Gouvernement dispose au total de vingt minutes pour intervenir.

La France a-t-elle un problème avec la police ? Le sujet des violences policières fait trop souvent l'actualité et la polémique a encore été alimentée ces derniers jours. Nous avons vu des images, qui, comme l'affirme le Président de la République, « nous font honte ». L'article 24 de la proposition de loi relative à la sécurité globale, qui sera bientôt soumise à l'examen de notre assemblée, cristallise une colère qui semble sur le point de se déchaîner. Ceux qui y voient un blanc-seing délivré aux forces de l'ordre profitent des récentes violences policières pour jeter l'opprobre sur l'ensemble de la profession, en accusant le Gouvernement de la soutenir, voire de la couvrir. Disons-le tout net : oui, il y a parmi les forces de l'ordre des fonctionnaires qui commettent des actes répréhensibles, sur lesquels la justice doit se prononcer. Cependant, il me semble que nous portons tous une partie de la responsabilité de ces images de la honte. Le métier des forces de l'ordre est dangereux. De nombreux agents sont blessés et tués chaque année. En première ligne dans le combat contre le terrorisme, ils continuent d'assumer leurs missions de maintien de l'ordre public et de lutte contre le crime. Ils s'usent à arrêter des délinquants aussi vite relâchés, qui ne se gênent pas pour les narguer. L'immense majorité d'entre eux accomplissent leurs fonctions avec l'exemplarité à laquelle ils sont astreints, risquant leur vie, parfois celle de leur famille. que leurs conditions de travail sont telles qu'environ 40 policiers et 30 gendarmes se suicident chaque année. Il n'est pas ici question de chercher des excuses à des comportements qui ne sauraient le justifier il s'agit de prendre conscience que les conditions de travail de nos forces de l'ordre ne contribuent pas suffisamment à garantir leur sécurité et celle de nos concitoyens. Nous devons remédier à cela si nous voulons aller vers une société plus apaisée. À cet égard, nous soutenons la poursuite du plan de recrutement. Le maintien de la paix durant les manifestations du mouvement des gilets jaunes a montré les limites d'un effectif insuffisant. La quantité d'heures supplémentaires non payées illustre aussi la nécessité d'un recrutement massif malgré les mesures prises, il en restait près de 22 millions au mois de juin dernier. Ce chiffre est colossal ; il dit beaucoup de la réalité du terrain et des limites du modèle actuel. La création de près de 1 500 postes pour l'année 2021 est donc la bienvenue. Il faudra veiller à ce que cette augmentation des effectifs serve à soulager les unités les plus exposées. Pas assez nombreux, nos gendarmes et nos policiers ne sont pas non plus assez équipés. Ce projet de loi de finances prévoit un effort significatif, tant pour renouveler le matériel des fonctionnaires que pour réhabiliter le parc immobilier. Une attention particulière a été portée aux flottes de véhicules de la police et de la gendarmerie. Le vieillissement est un problème qu'il faut rapidement résoudre et nous saluons le fait que le Gouvernement s'y attelle ce projet de loi de finances. Concernant l'équipement, nous voulons encourager le Gouvernement à investir davantage dans un matériel essentiel que notre groupe Les Indépendants soutient depuis longtemps, à savoir les caméras mobiles. Voilà plus de deux ans que la loi de Jean-Pierre Decool relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique a été votée et promulguée. Elle concerne les pompiers, les agents pénitentiaires, mais aussi les policiers. Nous regrettons que ces deux années n'aient pas été mieux employées pour avancer sur cette question. En effet, plusieurs études, dont certaines ont été conduites aux États-Unis, indiquent que le port de ces caméras par les policiers fait chuter significativement le nombre d'incidents liés à l'usage de la force, ainsi que le nombre de plaintes contre les policiers. Nous sommes convaincus que leur utilisation peut grandement contribuer à renforcer la sécurité des fonctionnaires et la confiance de nos concitoyens. Par ailleurs, le parc immobilier se trouve dans une situation préoccupante. La réponse apportée d'année en année au besoin de rénovation n'est pas suffisante. Le plan de relance remédiera y pour 2021, mais n'apporte pas de solution durable. Les moyens de la mission « Sécurités » progressent cette année encore. Le contexte sécuritaire et social rend ce renforcement d'autant plus nécessaire. Pour qu'elles puissent remplir leurs missions dans des conditions optimales, pour la sécurité de tous, nos forces de l'ordre ont besoin d'encore plus de moyens. Le budget 2021 participe à cette montée en puissance, mais nous souhaiterions qu'elle soit davantage pérennisée. L'État devra trouver les financements pour ce faire, car, si la qualité a un prix, le manque de moyens finit aussi par se payer tôt ou tard.

Monsieur le président, madame la ministre, mesdames, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, la mission « Sécurités », qui nous est aujourd'hui présentée, n'est pas exempte de défauts.

d'autant plus que les efforts de dépenses se concentrent sur les programmes concernant la police et la gendarmerie nationales, qui verront leurs effectifs augmenter respectivement de 1 145 et 317 postes. Nous accueillons également avec satisfaction les décisions gouvernementales permettant la revalorisation de 150 euros accordée aux 22 000 policiers travaillant de nuit, ou les 26,5 millions d'euros destinés au paiement de leurs heures supplémentaires. Les dépenses croissantes en matière d'équipements sont également positives, notamment dans le cadre du renouvellement des parcs automobiles des policiers et gendarmes. Enfin, nous notons avec intérêt l'achat de 21 000 caméras-piétons, qui peuvent être des outils favorisant l'exemplarité de nos forces de l'ordre dans l'exercice de leurs prérogatives, à condition, bien sûr, qu'elles fonctionnent. Tous les éléments visant à améliorer les conditions de travail, sociales et salariales de nos fonctionnaires de la sécurité intérieure doivent être salués. Cela n'est que justice, tant la profession est mise sous pression. Pourtant, il est à craindre que ces gages ne soient pas de nature à dissiper totalement le malaise qu'expriment régulièrement les gardiens de la paix. Depuis 2003 et la suppression de la police de proximité, les gouvernements successifs ont multiplié les décisions hasardeuses. Celles-ci ont fortement affecté les effectifs de la police nationale, notamment au cours du mandat de Nicolas Sarkozy, mais ont aussi eu pour effet délétère d'abîmer le lien entre la population française et les forces de l'ordre, régulièrement accusées de comportements violents, discriminatoires et arbitraires. La confiance doit donc être retrouvée entre la Nation française et sa police républicaine. Pour ce faire, une meilleure formation doit être offerte à nos policiers et gendarmes. Des fonctionnaires mieux formés sont des fonctionnaires qui optent pour des méthodes de maintien de l'ordre plus adaptées, qui reçoivent les plaintes de manière adéquate et qui nouent du lien social avec leurs concitoyens. Somme toute, un policier mieux formé est un policier qui protège mieux. Il est donc vital qu'à l'avenir la hausse des crédits destinés à la formation des forces de l'ordre soit le corollaire de l'ouverture

pour ces personnels. Je termine en mentionnant la situation du programme 161, « Sécurité civile ». Certains se satisferont peut-être de la maigre augmentation des crédits alloués, à hauteur de 0,45 %. Il n'en reste pas moins que ce programme ne représente que 7 % des dépenses réalisées en matière de sécurité civile, et que 90 % du financement de celle-ci pèse sur le budget des collectivités territoriales. Face aux changements climatiques et aux risques sanitaires et naturels que ces derniers sont susceptibles d'entraîner, il est vital que le concours de l'État se fasse plus important, afin de soutenir les localités face à ces périls du XXI siècle. L'ouverture de nouveaux postes dans la police et la gendarmerie, les renforcements des moyens des renseignements, ainsi que les investissements dans les équipements du ministère de l'intérieur sont de bonnes nouvelles, mais nous nous devons d'attirer l'attention de l'exécutif sur les carences et sous-dotations de ce budget, notamment en matière de formation et de sécurité civile. Pour ces raisons, les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s'abstiendront de voter les crédits de cette mission. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je profite de cette intervention pour rendre hommage à nos forces de l'ordre, qui vivent une année extrêmement éprouvante, avec une mobilisation sans faille sur tous les fronts. Sans sécurité, aucune liberté n'est pleinement effective. Aujourd'hui, il y a autant d'insécurités qu'il y a de situations pour les Français : ruralité, urbanité, dans le foyer ou en dehors, de la violence conjugale aux violences urbaines.

Aucun aspect n'a été oublié dans les programmes de ce budget pour 2021. Madame la ministre, vous voulez faire évoluer la répartition des tâches entre police et gendarmerie pour aller vers une organisation plus efficace. Vous avez, dans le même temps, insisté sur la nécessité de maintenir ces deux forces complémentaires, tout en ouvrant ce chantier, qui n'avait pas été touché depuis des dizaines d'années. Or les agglomérations se sont étendues géographiquement. Pour répondre aux nouveaux défis, l'idée est d'apporter des synergies dans les domaines qui exigent une action conjointe. Je pense notamment au maintien de l'ordre, mais aussi aux domaines de forte compétence, comme la police technique et scientifique ou le cyber. Indépendamment de la façon dont nous envisageons les rapports entre les forces de sécurité intérieure et les citoyens, il est essentiel que celles-ci soient bien recrutées, bien formées et bien équipées. Pour ce faire, un budget important est nécessaire. Pour l'année 2021, les crédits demandés pour la mission atteignent un montant de 21,23 milliards d'euros en autorisations d'engagement et de 20,7 milliards d'euros en crédits de paiement. Cela représente une hausse d'environ 1,05 % par rapport à la loi de finances initiale pour 2020. Lors de l'examen à l'Assemblée nationale, les crédits de la mission ont été majorés de 33,3 millions d'euros pour les dépenses de personnels, la hausse étant répartie sur les programmes « Police nationale

Il est également prévu un effort spécifique pour les services de renseignement et de lutte contre le terrorisme, avec 330 créations d'emplois supplémentaires. Ce budget pour 2021 poursuit ainsi pleinement la mise en oeuvre du plan de recrutement ambitieux de 10 000 policiers et gendarmes sur le quinquennat. Si ces dépenses de personnes peuvent être difficilement pilotables, le plan de relance vient, dans le même temps, renforcer l'effort pour « s'occuper du quotidien du policier et du gendarme » et assurer le plein maintien de leurs capacités opérationnelles. Si l'on inclut ce plan, l'augmentation des crédits de la mission s'élève à 621 millions d'euros en crédits de fonctionnement et à 455 millions d'euros en crédits d'investissement. Cela porte l'augmentation du budget de la mission « Sécurités » à 1,7 milliard d'euros Je salue la création d'une indemnité de travail de nuit pour la police nationale, le renouvellement du parc automobile de la police et de la gendarmerie, à hauteur de 213 millions d'euros, ainsi que la dotation complémentaire pour la généralisation de l'utilisation des caméras-piétons au mois de juillet 2021. Le budget est axé autour de trois priorités stratégiques, qui correspondent à trois grandes luttes nationales : contre les stupéfiants, contre les séparatismes et contre les violences conjugales. La police et la gendarmerie sont traitées équitablement. Le programme 176, « Police nationale » prévoit 11,14 milliards d'euros et le programme 152, « Gendarmerie nationale », 9 milliards L'objectif est d'évaluer la prévention et l'activité répressive des forces de sécurité et de renforcer l'activité des services pour mieux combattre la délinquance. Il faut aussi optimiser l'emploi des forces mobiles, renforcer l'efficacité dans la lutte contre l'insécurité routière, ainsi que la transparence du service public de sécurité intérieure. Un danger majeur concerne l'ensemble de nos concitoyens : la menace terroriste. Nous avons été plusieurs fois durement frappés récemment, jusqu'aux portes de nos écoles, jusqu'aux parvis des lieux de culte. Cette menace, qui est une priorité absolue, est bien prise en compte dans chacun des crédits de la mission. Il ne faut pas non plus négliger certains dangers du quotidien. Je pense à ceux qui surgissent au détour d'un simple trajet en voiture. Le programme 207, « Sécurité et éducation routières vise à mobiliser l'ensemble de la sécurité routière pour réduire le nombre d'accidents sur les routes et améliorer le service du permis de conduire ; il est appuyé par 41,2 millions d'euros. Enfin, il faut prendre en compte la prévention et la prédiction d'autres dangers, en appui sur les moyens des services départementaux d'incendie et de secours. Pour permettre à nos forces de répondre efficacement à ces dangers, le programme 161, « Sécurité civile » augmente de 2,3 millions d'euros, pour atteindre plus de 520 millions d'euros. d'euros. Madame la ministre, pourrez-vous préciser les dépenses pour la sécurité civile aujourd'hui inscrites dans plusieurs programmes qui n'entrent pas dans cette mission ? Pour finir, je salue le Livre blanc de la sécurité intérieure, dans lequel se retrouve l'ambition de ce budget pour 2021. Certaines de ses mesures, en matière notamment de sécurité privée et de police municipale, sont déclinées dans la proposition de loi relative à la sécurité globale. La Haute Assemblée en sera prochainement saisie elle saura exercer pleinement ses prérogatives pour travailler ces dispositions dans un esprit d'équilibre entre sécurités et libertés. Suivant les avis de l'ensemble des rapporteurs spéciaux et des rapporteurs pour avis, le groupe RDPI votera les crédits de la mission, les articles rattachés, ainsi que les crédits du compte d'affectation spéciale.

madame la ministre, mes chers collègues, chacun s'accordera à dire que les questions liées à la sécurité trouvent dans notre pays un écho de plus en plus important, trop souvent pour de mauvaises raisons. De trop nombreuses lois, décisions gouvernementales ou juridictionnelles intéressant le maintien de l'ordre public sous toutes ses formes amènent leur lot de polémiques, là où nous devrions rechercher le consensus républicain quant aux finalités et le débat démocratique dans les modalités. C'est le rôle d'ailleurs dévolu au Parlement, me semble-t-il, en tant que représentant de la Nation : discuter la loi en toute transparence et améliorer sa rédaction grâce à la navette parlementaire. La discussion budgétaire en fait pleinement partie, puisqu'il est coutume de dire que, derrière les chiffres, c'est une politique qui est menée. Aussi, à notre sens et c'est notre préoccupation, ce budget devrait traiter du lien de confiance entre les forces de l'ordre et les citoyens, socle fondamental de la légitimité de l'État

la terrifiante attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne, mais aussi les agressions devenues régulières de fonctionnaires de police durant les interpellations, comme la semaine dernière en Seine-et-Marne de l'autre, l'indignation suscitée par les images de l'évacuation de la place de la République, voilà quinze jours, ou encore par celles du véritable passage à tabac de Michel Zecler, la semaine dernière. Que révèle cette triste litanie ? Qu'entre violence policière et violence contre les policiers, il y a un va-et-vient quasi schizophrénique, l'expression d'un symptôme préoccupant pour la santé de notre État de droit, voire de la confiance de nos concitoyens envers l'État, à l'heure où le complotisme a pignon sur rue et n'a rien à envier aux superstitions d'antan. L'heure n'est pas à prendre parti pour un camp ou un autre : il faut trouver la voie de l'apaisement, dans le respect de la loi et de l'ordre public. Notre Nation ne doit pas s'enliser dans ce chemin insupportable qui fait que, chaque semaine, de nouveaux événements alimentent les chaînes d'information, boulimiques de polémiques, et font le lit des populismes qui n'attendent que de prospérer sur cette crise de confiance. Certes, nous pourrons bien nous rassurer en nous disant que les gendarmes ou les pompiers conservent une bonne image dans la population, mais rien n'est acquis. Nous le constatons tous les jours. Notre réponse doit donc être pensée et structurée pour le long terme. Face à cela, le budget que nous examinons apporte des premiers éléments de réponse. en 2021 la mise en oeuvre du plan de recrutement de 10 000 policiers et gendarmes sur le quinquennat, conformément à la loi de programmation, en prévoyant la création nette de 1 145 emplois dans la police nationale et de 335 emplois dans la gendarmerie nationale. Ces emplois supplémentaires devraient principalement venir renforcer les effectifs de sécurité publique. Nous nous réjouissons de cette évolution. Néanmoins, cette évolution ne dit pas tout. Les enjeux liés aux missions de sécurité ne tiennent pas qu'à une question d'effectifs. Une fois le nouveau personnel recruté, encore faut-il qu'il puisse effectuer ses tâches dans des conditions à la hauteur de leur importance. Garantir l'ordre public est d'abord une question de moyens. Les gendarmes et les policiers nous alertent constamment là-dessus : ils doivent disposer des matériels qui leur permettront d'assurer leur mission efficacement. La formation de nos forces de l'ordre est devenue un enjeu essentiel, en particulier au regard de l'évolution de notre doctrine du maintien de l'ordre et des techniques d'interpellation, sujet sur lequel Catherine Di Folco Le budget de la mission « Sécurités » apporte encore des réponses en prévoyant de financer la modernisation des équipements, d'élargir le parc automobile ou encore d'engager des travaux de rénovation immobilière. Là aussi, c'est un motif Enfin, s'agissant des questions liées à la sécurité civile, nous soulignerons la légère hausse d'effectifs qui est prévue. Cependant, les crédits de cette mission sont stables. Or cette stagnation peut se révéler inquiétante, lorsque l'on sait qu'une grande partie de la sécurité civile est assumée

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cette mission a ceci d'étonnant que l'augmentation importante de ses crédits est principalement liée au plan de relance, avec, pour base, des annonces gouvernementales aux données budgétaires non consolidées. qui, comme l'a relevé le rapporteur spécial, nuit non seulement à la lisibilité, mais aussi et surtout à la sincérité de l'information communiquée au Parlement. Ainsi, hors plan de relance, les crédits de paiement de cette mission passent de 19,9 milliards d'euros à 20,21 milliards d'euros,

Cette augmentation « exceptionnelle » satisfait les syndicats. Nous pouvons le comprendre et nous en féliciter, dans le sens où elle apporte des réponses à des questions récurrentes. de la revalorisation de 150 euros accordée aux 22 000 nuiteux, de la relance des discussions sur la gratuité des transports pour les policiers ou de la revalorisation des heures supplémentaires. Surtout, cela représente une occasion unique pour le ministère de l'intérieur de donner un coup d'arrêt à la dégradation des conditions de travail et de procéder à la remise à niveau des équipements. Reste l'effort est ponctuel et imputable à la crise sanitaire en cours. Or la situation matérielle dégradée de nos forces de l'ordre nécessite une réponse durable et une revalorisation pérenne des crédits de fonctionnement et d'investissement. Nos convergences avec la majorité sénatoriale sur cette mission s'arrêtent là En matière de sécurité publique, nos principales critiques ont toujours principalement porté sur la politique menée, donc budgétisée, qui pose de nombreuses difficultés.

Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de stigmatiser nos forces de l'ordre, qui sont confrontées au quotidien à la misère sociale et dont le travail anxiogène donne trop souvent lieu au pire. mal-être policier et violences policières, deux tabous de notre société, doivent être abordés avec la même rigueur et sans détour. L'actualité brûlante dans laquelle s'inscrit cette discussion nous y invite plus que jamais. Si l'attention médiatique s'est focalisée sur l'article 24 de la loi relative que nous pointons un autre problème d'envergure : le glissement dangereux de notre sécurité publique vers une privatisation. Il s'agit d'un enjeu phare qui n'aura pas échappé à la lecture de la commission des lois, puisque le rapporteur souhaite, pour alléger les tâches de procédure pénale, pour renforcer la présence policière dans l'espace public et diminuer leurs missions « périphériques », « la montée en puissance des autres acteurs de la sécurité », comme le suggère précisément ce texte à l'origine de la crise politique en cours et comme le ministre de l'intérieur l'appelle de ses voeux dans le Livre blanc de la Pour notre part, nous persistons à dire que la sécurité publique est du ressort du pouvoir régalien et que les fonctionnaires de police et de gendarmerie sont des acteurs du service public. Glisser vers une privatisation n'améliorera en rien les conditions de travail de nos forces de l'ordre. Vouloir se couper de la police républicaine au profit d'un service de sécurité mercantile et servile, bien éloigné des fonctions régaliennes de l'État, est une grave erreur. En réalité, cette question de la présence dans l'espace public de nos forces de l'ordre est non pas une question budgétaire, mais une question de doctrine d'emploi des forces de l'ordre. C'est une question éminemment politique ! Le chemin est encore long pour que convergent notre conception de la police républicaine et l'idée que vous vous en faites. C'est pourquoi nous voterons contre ces crédits, qui, d'ailleurs,

à l'occasion du débat sur les crédits de la mission « Sécurités », permettez-moi, tant en mon nom personnel qu'au nom de mon groupe, de marquer mon soutien

des Français. Jamais le climat social n'a été aussi tendu et jamais la demande d'ordre n'a été aussi multiple. De la sécurité des maires et des élus, en passant par celle des transports, la lutte contre les trafics et celle contre le terrorisme, la cybercriminalité, les débordements et violences des rues, les violences faites aux femmes, la demande de sécurité est polymorphe et urgente. Elle est aussi impérative, pour que notre pays ne glisse pas dans les bras extrêmes, qui encaissent les bénéfices des désordres que nous voyons trop souvent sur les chaînes d'information continue. Le dialogue a disparu de nos sociétés et fait place aux invectives relayées par les médias et les réseaux sociaux. La violence est un signe de mauvaise santé de notre société. Face à ce constat que chacun peut faire, il nous appartient de tenter d'apporter des solutions, l'ajustement du curseur n'est pas toujours facile. L'an dernier, notre débat se déroulait en pleine crise des gilets jaunes. La semaine dernière, des violences inadmissibles ont été commises contre des policiers,

Je ne doute pas qu'elle le soit dans son immense majorité, mais une petite minorité vient salir le travail et l'engagement de dizaines de milliers de fonctionnaires. L'inspection

Si la fonction de renseignement de l'IGPN ne semble pas devoir être critiquée, tel n'est pas le cas de sa mission de contrôle. Pendant l'année 2019, selon son dernier rapport, 1 460 enquêtes judiciaires ont été menées. Cette hausse est notamment due à la multiplication des mouvements sociaux.

lors, sans même être rendue indépendante du ministère de l'intérieur, l'IGPN pourrait comprendre un comité citoyen, ou d'autres membres de la société civile, ainsi que des magistrats et, pourquoi pas,

Faut-il revoir les critères d'évaluation de la police ? Doit-on, par exemple, modifier le régime de la charge de la preuve ou accroître la transparence ? de M. Christophe Naegelen sur la situation, les missions et les moyens des forces de sécurité, qu'il s'agisse de la police nationale, de la gendarmerie ou de la police municipale.

dès lors que les loyers sont payés, il faut que les collectivités locales puissent assurer l'hébergement des forces de sécurité et de leurs familles dans des conditions satisfaisantes. Le deuxième message concerne la gendarmerie de Tourouvre-au-Perche,

particulièrement dynamiques pour nos forces de maintien de l'ordre. Des jeunes sont prêts à vivre à 20 000 kilomètres de leur famille et de leurs amis pour défendre notre souveraineté et maintenir l'ordre public. Pourtant, ces agents du Pacifique sont à l'heure actuelle exclus cette prime spécifique d'installation, que touchent pourtant leurs collègues des autres territoires ultramarins affectés en métropole. Saisie de cette question par Gérard Poadja, Mme la ministre de la défense s'est engagée à traiter cette discrimination. J'espère, madame la ministre, que vous pourrez également soutenir cette démarche. Sous le bénéfice de ces

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les milices d'extrême gauche, relayées par certains parlementaires et éditorialistes, croient bon d'évoquer un « problème systémique » dans la police. S'il y a quelque chose de systémique, c'est bien la haine du flic chez ces gens-là et la violence des anarchistes dans nos rues ! De qui il parle ? Moi, je vous le dis tout net : je soutiens la police de toutes mes forces. Je soutiens nos policiers, comme ces hommes de la brigade anticriminalité (BAC) que j'ai accompagnés pendant toute une nuit dans les quartiers nord et le centre de Marseille ; ils faisaient ce qu'ils pouvaient, malgré les consignes non écrites de « ne pas faire de vagues », malgré l'équipement usé, malgré les effectifs réduits, malgré les provocations. Je veux rappeler ici aux Français que les forces de l'ordre sont prêtes à donner leur vie pour sauver la nôtre, comme les hommes qui ont abattu les terroristes de Nice et de Conflans-Sainte-Honorine, comme ceux qui sont entrés sous les balles dans le Bataclan, comme ceux qui sont morts sous les balles des frères Kouachi ou comme celui qui a neutralisé l'assassin de Laura et Mauranne à Marseille. On voudrait nous faire croire que les Français ne soutiennent pas leur police ; rien n'est plus faux ! Connaissez-vous un seul Français qui ait déménagé parce qu'un commissariat ouvrait près de chez lui ? Madame la ministre, je ne ferai pas porter le chapeau à votre seul gouvernement de l'état des équipements et du moral des policiers ils sont le résultat de décennies d'inaction gouvernementale. Seulement, la situation empire ! Nos forces de sécurité sont sollicitées en permanence et elles n'en peuvent plus. Elles sont pourtant le dernier rempart avant le chaos.

nécessaires pour payer les 24 millions d'heures supplémentaires effectuées. Vous affirmez vouloir faire un effort de 63 millions d'euros, soit quatre fois moins que nécessaire. Ce que demande avant tout la police, c'est de pouvoir travailler dans de bonnes conditions et d'être respectée par ceux qui la dirigent. Quand l'ancien ministre de l'intérieur a envisagé d'organiser une cérémonie, place Beauvau, où des policiers mettraient un genou à terre, c'était de l'humiliation ! Quand un Président de la République en fonction se met en scène au chevet d'une victime supposée qui accuse des policiers de violences, et ce avant toute enquête, c'est une humiliation Quand l'actuel ministre de la justice affirmait, il y a quelques mois, dans l'affaire Théo, que la police devait présenter des excuses, comment voulez-vous que celle-ci ait confiance en lui ? La police ne croit plus en ses chefs. Elle ne croit plus en son ministre. Elle dont l'offensive sécuritaire s'est dégonflée sous le poids de la rue conquise et saccagée par 10 000 manifestants d'extrême gauche ! Elle ne croit plus en lui, qui a demandé la révocation de policiers qui sont déjà derrière les barreaux sans même avoir été entendus, pendant que la racaille multirécidiviste sort libre des commissariats faute de place en prison Le ministre de l'intérieur a lâché ses hommes ; ils ne l'oublieront pas ! Mal payées, mal équipées, mal dirigées, mal considérées : voilà le quotidien de nos forces de l'ordre. Quant à moi, je ne lâche pas ces gendarmes et ces policiers nationaux et municipaux, mais je leur dis : Comme moi, le pays réel vous soutient. Tenez bon ! Bientôt, nous allons remettre la France en ordre

ma part, madame la ministre, vous interpeller sur des sujets de sécurité civile que vous connaissez. Ces enjeux sont importants pour le quotidien des 41 000 sapeurs-pompiers professionnels et des 198 000 sapeurs-pompiers volontaires. ces derniers représentent 79 % des sapeurs-pompiers de France. Dans mon département de l'Indre, comme dans de nombreux départements ruraux, ils réalisent la grande majorité des interventions. Sans ces femmes et ces hommes qui donnent de leur temps au péril de leur vie, beaucoup de nos campagnes n'auraient quasiment plus de secours. Aujourd'hui- et c'est notamment la conséquence des

Comme vous le savez, madame la ministre, les pompiers se substituent aux transporteurs sanitaires privés pour des interventions non urgentes.

Il formule dix recommandations pour améliorer les pratiques, trop disparates selon les territoires, pour rationaliser le recours aux services de secours et d'incendie, pour assouplir les contraintes opérationnelles et pour revoir le fameux mode de calcul du tarif de l'indemnisation.

C'est une avancée considérable, surtout compte tenu des perspectives budgétaires des départements, mais elle ne compense pas totalement cette augmentation. En revanche, au-delà du parallélisme des formes, nous regrettons, madame la ministre, l'opposition du Gouvernement à la suppression de la part salariale de cette surcotisation.

ne remettre en cause ni le principe du volontariat ni le modèle français de sécurité civile, elle rappelle que c'est au cas par cas qu'elle se prononce, et non sur des organisations générales qui ne sont pas de sa compétence. Selon les critères retenus par l'Union européenne, c'est sur le caractère accessoire des revenus et de l'activité que l'attention doit être portée afin d'exonérer le volontariat du statut de travailleur.

pour donner le goût du volontariat à la population, à l'image des 29 000 jeunes sapeurs-pompiers, qui sont un bel exemple pour notre jeunesse. La parole

En traitant de ces crédits, nous aurons aussi à l'esprit les questions d'organisation de nos forces de sécurité, de commandement, d'encadrement, de déontologie et de doctrine d'emploi.

Pouvez-vous nous donner des indications sur les conséquences du choix d'une transmission dématérialisée, un que l'on espère souverain, des images enregistrées par les caméras-piétons ? ? Par ailleurs, une question se pose quant à l'effectivité du droit des citoyens à avoir accès aux images qui sont enregistrées d'eux. Si je ne me trompe, pour les caméras fixes, l'accès est supposé être direct. Or on a vu, dans l'histoire du jeune homme agressé au bois de Boulogne, que ce droit pouvait se révéler virtuel.

On a beaucoup parlé de la nécessité d'améliorer la formation initiale et continue des forces de l'ordre pour contribuer à la nécessaire réconciliation de la police avec la population. Nous avons donc déposé des amendements dans ce sens.

Cette année, un élément supplémentaire est venu s'ajouter : le financement de l'État en faveur de la sécurité civile devient de moins en moins lisible, sachant qu'il repose désormais sur dix programmes, pilotés par six ministères différents. Le programme 161 ne représentera plus en 2021 que 43 % de l'effort financier de l'État pour la sécurité civile, contre 50 % ces dernières années. Notre attention doit aussi se porter sur la situation financière des associations agréées pendant une crise sanitaire qui met à mal leur trésorerie. Le soutien de l'État se révèle nécessaire, faute de quoi elles risquent de ne plus pouvoir poursuivre leurs actions, qui sont unanimement reconnues, aux côtés des sapeurs-pompiers. Acteurs essentiels de la sécurité civile, ces derniers ont, entre le mois de mars et le mois de mai 2020, effectué plus de 122 000 interventions de secours d'urgence afin de porter assistance à des personnes présentant des symptômes de la covid-19, le plus souvent pour les transporter vers un centre hospitalier. La question des carences ambulancières est rapidement abordée quand on a l'occasion d'échanger avec un officier des SDIS. Ce sujet appelle, sur le terrain, une meilleure collaboration entre les SDIS et les services d'aide médicale urgente

Dès lors que le Gouvernement a reconnu l'existence de problèmes systémiques, nous devons tous travailler à pacifier les relations entre la police de la République et les citoyens. Il ne faudrait pas que ces problèmes systémiques et les égarements de quelques-uns nous fassent oublier la vertu du plus grand nombre. Les réformes, les clarifications et les modernisations doivent désormais venir vite, madame la ministre. C'est le sens de nos apports à cette construction budgétaire.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, la sécurité est devenue l'une des premières préoccupations des Français. Ces derniers mois ont vu le modèle républicain de sécurité durement mis à l'épreuve. Nouvelles attaques terroristes, persistance des radicalismes de tous bords, augmentation préoccupante des atteintes aux personnes, catastrophes naturelles telles que la tempête Alex : les défis à relever étaient innombrables. L'examen du budget de la mission « Sécurités » nous permet d'abord d'évaluer l'adéquation des moyens prévus avec l'ampleur de ces défis. À cet égard, nous constatons un effort d'investissement important, grâce au plan de relance. Nous nous en félicitons. Au-delà de cette réponse ponctuelle, décidée dans le cadre de la crise sanitaire, il est toutefois nécessaire d'anticiper les défis du jour d'après. Le nouveau Livre blanc de la sécurité intérieure permet précisément de se livrer à cet exercice. Il doit également constituer la matrice d'une future loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure

Or cette singularité des gendarmes est pourtant un aspect central du modèle de sécurité intérieure français, que le rattachement des gendarmes au ministère de l'intérieur en 2009 n'a pas remis en cause. La réactivité de la gendarmerie nationale, sa polyvalence et sa capacité à répondre présent auprès des populations et des élus en toutes circonstances, le tout dans le respect des règles républicaines, découlent en grande partie de ce statut militaire. C'est bien lui qui garantit la résilience et la disponibilité de la gendarmerie nationale. Aussi, nous sommes très attachés à ce modèle. C'est pourquoi il ne faut en aucun cas le laisser se scléroser. Cela suppose, en premier lieu, de reconnaître les sujétions imposées par l'état militaire et de prendre les mesures de ressources humaines et d'investissement qui en sont la contrepartie nécessaire. Contrairement aux policiers, les gendarmes ne peuvent pas se syndiquer, même si nous avons approuvé, en 2015, la création des associations professionnelles nationales de militaires (APNM), qui ont ouvert des possibilités limitées de revendication. C'est donc le rôle de la représentation nationale que d'évaluer constamment le respect de l'équilibre entre les sujétions liées à la condition militaire et les mesures dont bénéficient les gendarmes. les gendarmes. Les mutualisations avec la police nationale, qui sont nécessaires et utiles dans le domaine des fonctions de support ou de la police technique et scientifique, ne doivent pas porter atteinte à la spécificité du statut des gendarmes ni aux domaines d'excellence de la gendarmerie. Nous nous étions ainsi émus, l'année dernière, des projets de centralisation ministérielle des fonctions liées au numérique. Par chance, nous avons été entendus et la gendarmerie a pu continuer à innover dans ce domaine. Par ailleurs, la gendarmerie ne peut rester à l'écart des débats sur l'équilibre nécessaire entre sécurités et libertés. Ainsi, dans le domaine du maintien de l'ordre, la doctrine doit être modernisée en permanence. C'est aussi le cas pour l'utilisation des technologies numériques. Les drones, la généralisation des caméras-piétons ou encore la numérisation intégrale des procédures suscitent des interrogations et des réticences, comme l'a montré le débat autour de l'application GendNotes. Nous avons une totale confiance dans la capacité de la gendarmerie à relever ces défis. En effet, le statut militaire, loin d'être un handicap, constitue selon nous un atout dans cet exercice délicat de conciliation entre éthique républicaine et sécurité. Comme la commission d'enquête du Sénat sur l'état des forces de sécurité intérieure l'a déjà établi il y a deux ans, la police nationale connaît actuellement une crise multifactorielle. Ne croyons pas que la gendarmerie soit à l'abri de telles vicissitudes ! Au contraire, l'histoire nous invite à la prudence. À nous et à vous, madame la ministre, de faire évoluer ce modèle et de l'améliorer constamment, afin qu'il continue à offrir un service de sécurité de proximité unanimement apprécié

il vous revient d'examiner les crédits inscrits au projet de loi de finances pour 2021 au titre de trois missions budgétaires, relevant du ministère de l'intérieur, en commençant par la mission « Sécurités » et le compte d'affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ». Comme le ministre de l'intérieur et moi-même l'avons fait, voilà quelques jours, devant la commission des lois, je veux tout d'abord me réjouir que, conformément à la volonté du Président de la République et du Premier ministre, le budget du ministère de l'intérieur connaisse une augmentation significative de ses crédits, de 1,14 milliard d'euros. Cette augmentation des crédits est rendue possible tant par l'augmentation du budget dit « ordinaire », à hauteur de 400 millions d'euros, que par un premier renfort du plan de relance, à hauteur de 740 millions d'euros, hors appels à projets.

La première de ces priorités est d'imposer les valeurs de la République sur l'ensemble du territoire national. Au cours des dernières années, notre pays a de plus en plus souvent été l'objet d'attaques de la part de groupes organisés, notamment liés à l'islamisme radical. À cet égard, le projet de loi confortant les principes républicains sera déposé dans quelques jours. Notre deuxième priorité est de mener une lutte intense contre les stupéfiants, qui sont à l'origine de nombreux faits de délinquance, de l'insécurité du quotidien jusqu'aux règlements de compte les plus violents, en passant par le narcobanditisme et le financement du terrorisme. Notre troisième priorité, enfin, est de lutter contre les violences conjugales, sexistes et sexuelles. Le Président de la République en a fait la grande cause du quinquennat. Nous devons agir sans relâche en continuant le travail d'accueil des victimes de ces violences et en apportant des réponses immédiates et fortes à ces faits. À cet égard, le ministère de l'intérieur est le premier contributeur, en moyens tant humains que financiers, à la protection des femmes

singulièrement des forces de sécurité, afin de donner à nos agents les moyens d'agir et d'exercer leur métier dans des conditions dignes. Ainsi, cette année, les crédits de la mission « Sécurités » sont en forte augmentation : en prenant en considération le plan France Relance, la progression des crédits est de 645 millions d'euros

de ce dernier poste, je tiens à indiquer à la représentation nationale que, grâce aux crédits adoptés par les parlementaires, nous pourrons engager, d'ici à la fin de l'année, plus de 5 000 opérations, pour 26 millions d'euros, dans nos casernes de gendarmerie

à la sécurité civile, notre objectif est de renforcer sa capacité de prévention, d'anticipation et d'adaptation. C'est une nécessité pour faire face aux événements et aux catastrophes naturelles, comme nous l'a encore, hélas, démontré la tempête Alex, qui a durement frappé les Alpes-Maritimes le 2 octobre dernier. Au titre du seul programme 161, les crédits

entre 2018 et 2020. Cette pratique se poursuivra dans quatre nouvelles régions- Hauts-de-France, Grand Est, Nouvelle-Aquitaine, Bourgogne-Franche-Comté -, avant d'être progressivement étendue à de nouvelles régions métropolitaines.